pour dénoncer le manque de postes, les conditions de travail intolérables, les budgets indignes. Fait exceptionnel, cet appel à la mobilisation était lancé par l'ensemble des organisations, les syndicats comme les structures représentatives des directeurs des établissements d'aide à la personne. Toutes et tous dénoncent la maltraitance institutionnelle qui touche à la fois les personnels- une majorité de femmes, précaires, mal payées -et les personnes dont ils ont la charge. Mon collègue Dominique Watrin vous a interpellée, à maintes reprises, sur ce sujet.

au sein de notre société, qui leur donne vraiment une place à part entière parmi nous. Je rappelle que nous allons passer de 1,5 million de personnes âgées de plus de 85 ans à 5 millions en 2050. L'État assume. L'État s'engage dans cette évolution du grand âge. Nous augmentons les crédits alloués aux soins de plus de 400 millions d'euros. Je rappelle que, sur la partie « soins », le financement de la sécurité sociale est passé de 5 à 10 milliards d'euros entre 2007 et 2017. Au total, pour cette année, ce sont 160 millions d'euros supplémentaires que nous allons allouer aux EHPAD : 72 millions d'euros pour recruter du personnel et améliorer les prises en charge ; 10 millions d'euros pour recruter des infirmières de nuit 28 millions d'euros supplémentaires pour accompagner les EHPAD en difficulté ; enfin, j'ai débloqué, c'est exact, 50 millions d'euros supplémentaires pour appuyer ponctuellement les EHPAD, notamment publics, qui rencontrent le plus de difficultés dans les régions. Je rappelle que le modèle de financement est complexe. Il concerne l'État, les départements et les usagers. L'État a en charge la partie « soins ». En quelques années, les résidents accueillis en EHPAD sont de plus en plus dépendants, car ils restent plus longtemps à domicile. rend le travail des aides-soignants plus difficile, elle pose la question de la médicalisation et de l'importance du travail avec les médecins coordonnateurs et les infirmiers. La partie « dépendance » est assumée par les départements, il est primordial de travailler sur la dépendance, main dans la main, avec l'ensemble des présidents des conseils départementaux et des fédérations hospitalières, afin d'assurer l'évolution de notre système face à l'augmentation du nombre de personnes âgées dépendantes. La parole Madame la ministre, vous ne répondez pas au caractère d'urgence de la situation que vivent aussi bien des personnels que des résidents. La réforme de financement des EHPAD va pénaliser les établissements publics et non lucratifs, qui accueillent le plus grand nombre de personnes en difficulté.

Avec l'arrivée des fiches de paye de janvier, on assiste à un grand exercice d'autosatisfaction de la part du Gouvernement. Reprenant l'argumentaire d'Emmanuel Macron lorsqu'il était candidat à la présidentielle, vous-même, monsieur le secrétaire d'État, répétez à l'envi que vos mesures fiscales redonneraient du pouvoir d'achat à tous les Français. Pourtant, une étude récente de l'INSEE prévoit une perte de pouvoir d'achat pour nos concitoyens, notamment au premier trimestre de 2018. Avant de profiter d'une potentielle baisse de leur taxe d'habitation, ces derniers vont, en effet, voir leur pouvoir d'achat amputé de 0,7 point par rapport au dernier trimestre 2017. Et globalement, en 2018, il va diminuer de 0,3 % par rapport à l'an dernier. Surtout, sur cette question du pouvoir d'achat, force est de constater que la situation n'est pas la même pour tous. Les quelque 5,4 millions d'agents de la fonction publique ont, quant parfaitement compris que le fait de toucher une indemnité compensatrice du 1,7 point de hausse de CSG ne signifiait pas un gain de pouvoir d'achat. Rétablissement du jour de carence, gel de la valeur du point d'indice, report d'un an de l'accord « Parcours professionnels, carrières et rémunérations sans compter l'augmentation du coût de la vie en général, à la pompe, aux péages et sur la facture de gaz ... Tout cela va plutôt dans le sens d'un appauvrissement. Le malaise est palpable, comme le révèlent les mouvements observés récemment dans les prisons, les hôpitaux ou les EHPAD. Et que dire des retraités, autres victimes de la réforme fiscale ? Dans la vraie vie, de nombreux retraités ont de plus en plus de difficultés à payer certains actes médicaux, à disposer d'une mutuelle santé ou encore à s'acquitter de leurs dépenses d'énergie. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous dire ce que le Gouvernement compte mettre en oeuvre pour que tous les Français, et pas seulement les plus aisés, voient leur pouvoir d'achat augmenter ?

l'essentiel de votre question, si je l'ai bien comprise, portait sur la manière dont la hausse de la CSG est compensée pour les fonctionnaires, et plus généralement, ensuite, sur l'évolution du pouvoir d'achat des Français. votre question sur l'augmentation de la CSG, qui concerne les fonctionnaires comme l'ensemble des Français, il faut répéter, encore et toujours, que cette compensation est intégrale. Elle est intégrale, parce que nous avons supprimé la contribution de solidarité, la CES, pour celles et ceux qui y sont assujettis, c'est-à-dire celles et ceux qui ont un traitement brut de base supérieur à l'indice 313 en 2017. Elle est intégrale, puisque l'État a provisionné presque 300 millions d'euros pour verser une indemnité compensatrice aux agents publics, de manière que cette compensation soit parfaite et à l'euro près. Elle est intégrale, enfin, puisque l'État, de la même manière, a publié un décret, le 31 décembre dernier, pour abaisser le taux de cotisation maladie des employeurs publics de 11,5 % à 9,8 %, afin que les collectivités locales et les établissements hospitaliers puissent dégager les marges de manoeuvre nécessaires à cette compensation intégrale. Il faut le souligner et saluer les efforts de l'administration pour mettre à jour

avec la cotisation du secteur privé. J'en viens à la question du pouvoir d'achat. Nous pourrions, madame la sénatrice, nous rejoindre sur un certain nombre de mesures qui ont été prises par le Gouvernement et que vous retrouvez dans le projet de loi de finances pour 2018 : l'augmentation du minimum vieillesse, l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, le dégrèvement de la taxe d'habitation, à hauteur de 30 % pour 80 % des Français en 2018 et à hauteur de 100 % d'ici à 2020. Il y a quantité de mesures qui permettent, madame la sénatrice, à l'ensemble de nos concitoyens de voir leur pouvoir d'achat progresser. Le retour de la croissance viendra certainement contrecarrer les conclusions de l'étude que vous avez citée et dont certains aspects tiennent compte d'éléments extérieurs aux décisions du Gouvernement.

Monsieur le ministre d'État, ministre de l'intérieur, après le printemps 2016 qui a causé dans les esprits des sinistrés un réel traumatisme, plusieurs départements subissent à nouveau un épisode de crues dévastatrices. Ce sont au total 133 communes, pour la seule Seine-et-Marne, qui sont touchées par les inondations. Certaines, comme Condé-Sainte-Libiaire, qui connaîtra sa quatrième demande de classement en catastrophe naturelle depuis juin 2016, Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, est venu constater l'ampleur des dégâts lundi dernier à Saint-Mammès, Champagne-sur-Seine et Thomery, des communes lourdement affectées par la crue de la Seine et du Loing. Il faut imaginer la même désolation autour de l'Yonne, de l'Yerres, de la Marne, du Petit et du Grand Morin. Des maisons, des écoles, des commerces et des entreprises sont inondés, laissant les sinistrés dans le plus grand désarroi. Dans quelques jours, nous le souhaitons tous vivement, l'heure sera enfin à la décrue, à l'évaluation des dégâts et aux réparations. Monsieur le ministre, il y a urgence : urgence à déclarer les territoires touchés en état de catastrophe naturelle, urgence à mobiliser les assureurs pour qu'ils puissent, dans un premier temps, accorder des avances aux sinistrés, sachant que le montant des franchises pour les communes et les commerçants est important et que les primes d'assurance ont augmenté pour nombre d'assurés.

Monsieur le ministre, la solidarité dans les communes est exemplaire. Les maires et leurs équipes, dont la mobilisation est totale pour porter secours et organiser l'accueil des citoyens sinistrés, comme celle des pompiers et de la sécurité civile, comptent sur le soutien financier de l'État pour remettre en service les infrastructures publiques endommagées. Pouvez-vous donc nous dire quel sera l'engagement de l'État pour répondre à ces défis, malheureusement récurrents, que nous lance la nature

Le secteur de Nemours et les bords du Loing n'ont heureusement pas revécu, à ce jour, la situation qu'ils avaient connue il y a deux ans. Néanmoins, vous avez raison les dégâts sont extrêmement importants. Je partage donc pleinement votre volonté d'assurer, pour les victimes de ces inondations, une instruction très rapide des demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

le Gouvernement s'engage à réunir la commission de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle en procédure accélérée, avant même le constat de l'intégralité des dégâts. Je tiens également à préciser que les dégâts d'infrastructure ou de voirie qui pourraient être constatés relèvent de la procédure d'indemnisation des collectivités locales au titre de la dotation de solidarité pour événements climatiques et géologiques. Ce dispositif est doté, cette année, de 39 millions

Du fait du niveau de dépendance de ces résidents, du fait, en conséquence, de l'aggravation de leurs problèmes médicaux et du fait de l'augmentation des troubles du comportement, les besoins de soins et de soutien aux résidents des EHPAD sont croissants. face à ces besoins croissants, les établissements sont confrontés à des manques de crédits alarmants. Le budget « soins » des établissements n'est pas alloué à l00 % ; avec la convergence, il faudra sept ans pour atteindre le plafond. Comment soigner dans ces conditions ? Le budget « dépendance », qui est calculé, depuis la réforme tarifaire mise en oeuvre au début de 2017, comme le budget « soins », a mis en évidence une baisse du tarif « dépendance » pour les établissements publics. Le budget « hébergement

la réforme tarifaire, dont l'impact à terme a été évalué à près de 200 millions d'euros de pertes pour les EHPAD publics. Dans ces circonstances, le désespoir touche les personnels, les familles et les directeurs d'EHPAD. Que comptez-vous faire, madame la ministre, pour améliorer dans l'avenir cette situation qui devient catastrophique ?

a augmenté grâce à un maintien à domicile qui s'est révélé efficace. Nous allons nommer un médiateur dans les prochains jours : M. Pierre Ricordeau, inspecteur général des affaires sociales, facilitera le dialogue entre l'administration et les fédérations hospitalières, afin de permettre un débat public serein

afin de prévenir l'absentéisme et de permettre à ces employeurs de prendre les mesures nécessaires concernant les conditions de travail. Cette étude a lieu dans les entreprises d'au moins 200 salariés, afin de rassurer le public quant à l'anonymat des données transmises.

Que l'on ne se méprenne pas : je n'entends faire ni le procès des employeurs ni celui de la CPAM. Le sujet est bien celui du bon usage des données de santé des citoyens. Madame la ministre, avant tout, j'en appelle à votre vigilance : êtes-vous prête à remettre en place les garde-fous nécessaires dans cette expérimentation qui échappe aux procédures habituelles ? par ailleurs, que le rôle de la CPAM soit de travailler sur ces sujets directement avec l'employeur, en s'exonérant du filtre du médecin du travail ? Doit-on y voir la remise en question de la médecine du travail elle-même ? Je n'ose y croire. La parole

de rappeler que, dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels, l'assurance maladie peut mener des actions ciblées auprès de ses différents publics, c'est-à-dire des professionnels de santé, des assurés salariés, mais aussi des employeurs. Depuis maintenant quelques années, nous observons une augmentation de l'incidence de pathologies pouvant avoir eu une origine professionnelle : lombalgies, troubles musculo-squelettiques ou encore troubles psychosociaux. Aussi l'assurance maladie a-t-elle décidé de mener une expérimentation en direction des grandes entreprises, pour les alerter sur leur prévention des risques. La démarche consiste à sensibiliser ces entreprises sur les motifs d'arrêt maladie, afin, d'une part, de les inciter à prendre toutes les mesures et les moyens de prévention nécessaires à la bonne santé de leurs salariés, et, d'autre part, de lutter contre l'absentéisme. Cette démarche respecte le secret médical et la réglementation concernant la protection des données de santé. À ce titre, pour répondre à vos interrogations, madame la sénatrice, le traitement de ces données est autorisé par le code de la sécurité sociale. En effet, les données statistiques partagées avec l'entreprise sont totalement anonymes et ne concernent que les entreprises de plus de 200 salariés, afin que le lien entre les causes d'absence et les salariés soit totalement impossible. À ce stade, l'expérimentation porte sur cinq entreprises seulement. Il n'est nullement question de remettre en doute la médecine du travail et son action, bien au contraire. Je veux redire ici mon attachement à une meilleure prévention des risques. Cette expérimentation va dans le sens de la protection des salariés, et non dans celui de la dénonciation. Je pense que, tout comme moi, madame la sénatrice, vous approuverez cette politique, qui vise à prévenir les risques pour mieux guérir, tout en respectant l'anonymat dans l'usage des données de santé. La parole

Je me fais aujourd'hui l'écho des troubles observés dans mon département à l'occasion de ce nouveau report, qui a suscité la grogne des syndicats de salariés et de patrons de Mayotte, lesquels ont décidé, en réaction, de ne pas désigner d'assesseurs au tribunal du travail, en remplacement de ceux dont les mandats expiraient Cette décision a conduit le président de cette juridiction à siéger seul, depuis le 1 janvier 2018, afin d'éviter la paralysie du tribunal et le renvoi des affaires Vous conviendrez, madame la garde des sceaux, que cette solution n'est à l'évidence pas satisfaisante, puisqu'elle soustrait la justice prud'homale à l'appréciation des représentants des salariés et des employeurs. Une fois de plus, les citoyens mahorais ont le sentiment d'être laissés pour compte. leurs attentes, madame la garde des sceaux, et que comptez-vous faire pour assurer la continuité du service public prud'homal à Mayotte dans les mêmes conditions que sur le reste du territoire ?

je vous remercie de votre question, qui me donne l'occasion de rappeler l'attention que le Gouvernement porte en permanence à nos concitoyens ultramarins et, en l'espèce, aux justiciables du département de Mayotte.

la première présidente de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion aurait été obligée de constater cette carence et de désigner un juge du tribunal de grande instance pour juger le contentieux du travail. Non seulement il n'y aurait donc pas eu de conseil des prud'hommes au 1 janvier 2018, mais Mayotte aurait également perdu son tribunal du travail. Je ne l'ai pas voulu, et je ne pense pas que ce soit non plus le souhait de ceux qui, parmi les partenaires sociaux, expriment aujourd'hui leur mécontentement. Notre volonté est bien plutôt de mettre à profit ce délai pour élaborer l'architecture d'un conseil des prud'hommes qui prenne en compte les spécificités locales et qui permette le recrutement d'un personnel formé dans le cadre des dispositions du code du travail actuellement applicables à Mayotte. Pour cela, une commission interministérielle a été créée ; elle se rendra à Mayotte pour mettre en place ces solutions.

cas, je ferais tout pour que la continuité du service public de la justice soit réellement opérationnelle à Mayotte, dans l'intérêt des justiciables. La parole

de fait, de déni de justice à Mayotte du fait de cette crise. Je vous sais gré de rester vigilante, pour que la justice puisse continuer de s'exercer dans ce département comme partout ailleurs dans la République.

lundi 22 janvier dernier, je me suis rendu au centre de détention de Lille-Annoeullin, à la demande des syndicats de fonctionnaires pénitentiaires. Alors que je discutais avec les fonctionnaires grévistes, j'ai été délogé, comme eux, par vos gendarmes mobiles, monsieur le ministre de l'intérieur. Je tiens à vous rassurer : je vais bien. Vos gendarmes ont été exceptionnellement gentils

Ces équipes, créées en 2015, assurent des missions à l'intérieur de l'établissement- fouilles, contrôles, déplacement de détenus -, mais aussi à l'extérieur du bâtiment ; c'est là qu'est le problème. Ces équipes déplorent l'inadaptation des moyens dont elles disposent, sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif, qu'il s'agisse de leurs

de pasticher Coluche, mes chers collègues : « Excusez-moi de vous déranger, mais pourriez-vous, s'il vous plaît, décliner votre identité ? Accepteriez-vous d'être fouillés ? Encore une fois, mille pardons de vous importuner ! » Bref, ces équipes n'ont aucun pouvoir à l'extérieur ! Madame la garde des sceaux, pour que l'action des ELAC soit plus efficace et déterminante pour la sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur des prisons,

pour pouvoir faire bénéficier les ELSP, très rapidement, de ces nouveaux équipements. J'estime que l'ensemble de ces dispositifs contribuera à renforcer la sécurité dans les établissements pénitentiaires, ce qui était la première demande des organisations représentatives des surveillants des établissements pénitentiaires.

... Pendant que vous étiez au pouvoir, je travaillais dans des établissements de santé, et j'aurais aimé que ces problèmes soient anticipés ! Mais je vais tout de même vous répondre. Nous avons anticipé dès notre arrivée au pouvoir, en constatant la dégradation de la situation dans les EHPAD. Nous avons effectivement alloué des moyens nécessaires aux soins. Nous avons renforcé les postes d'infirmières de nuit. Nous allons équiper tous les EHPAD en télémédecine. Nous avons évidemment

ma part, je voudrais rendre hommage à ce qui a été fait par le gouvernement précédent ! En effet, ce sont 700 millions d'euros qui ont sur la table pour

Le cap défini par le Premier ministre le 17 janvier dernier repose sur trois principes. C'est, premièrement, le retour de l'État de droit sur la zone de Notre-Dame-des-Landes, sur lequel nous ne ferons aucune concession, mais que nous souhaitons obtenir de la manière la plus apaisée possible. Le second principe est la médiation avec l'ensemble des acteurs de la région,

Comme nous nous y étions engagés, la RD 281, dite « route des chicanes », a été dégagée. Quant aux terres obstruées par les zadistes depuis 2012, le conseil départemental a commencé les travaux.

Comme vous le savez, le Sénat a constitué un groupe de travail sur le sujet, groupe auquel j'aurai plaisir à participer. J'ai d'ailleurs un plutôt favorable sur cette mesure. Si l'objectif de diminuer le nombre de morts sur ces portions de routes accidentogènes est louable,

ailleurs, il semblerait que la direction de la sécurité routière n'ait pas souhaité participer aux travaux des assises, alors qu'elle y a été conviée par le groupe d'experts. On ne peut que s'en étonner et le regretter Ma demande est donc double. Tout d'abord, pourquoi la sécurité routière n'a-t-elle pas participé aux Assises de la Mobilité ? Ensuite, et surtout, monsieur le Premier ministre, pouvez-vous attendre les conclusions du groupe de travail sénatorial avant de confirmer votre décision de modifier la réglementation ? Permettez-moi enfin un petit clin d'oeil. Dans son discours de voeux de ce mardi, le Président de la République a longuement insisté sur l'importance des évaluations dans le cadre de l'action publique. Il serait tout de même paradoxal que son gouvernement ne respecte pas cette ligne de conduite ! Je vous remercie,

Dans le Rhône, votre département, madame la sénatrice, au cours de l'année 2017, quelque 58 personnes ont trouvé la mort et 2 735 ont été blessées.

dans le cadre d'un plan, grâce auquel seront sanctionnées beaucoup plus lourdement la conduite en état d'ivresse, l'utilisation du téléphone portable en conduisant, la conduite sans permis de conduire, la conduite

tous les spécialistes en la matière. Vous imaginez bien, madame la sénatrice, qu'avant de prendre une décision dont je sais qu'elle est impopulaire, ne recherchant pas spécifiquement et spontanément l'impopularité, je me suis demandé si elle pouvait avoir un effet et j'ai interrogé les sachants,

La profession agricole s'inquiète fortement des propositions de nouveaux zonages. À lui seul, mon département représente quelque 40 % des communes non classées de la région Occitanie, alors que, en termes de revenus agricoles, il est classé au rang national, sur 93, et possède un potentiel agronomique parmi les plus faibles. Ces zones défavorisées ne sont pas juste dessinées sur une carte pour Bruxelles. Elles représentent une réalité physique, économique, sociale et, surtout, humaine. Si le zonage, tel que vous le proposez aujourd'hui, devait être maintenu, les départements de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Lot et bien d'autres verront verront leur biodiversité irrémédiablement bouleversée. En effet, nombre d'éleveurs et de jeunes agriculteurs cesseront leur activité. Pourtant, comme l'a souligné le président Macron lors de ses voeux le 25 janvier dernier, l'agriculture française a du talent et de la ténacité. Voilà qui me laisse à penser, monsieur le ministre, que la mobilisation des manifestants dans nos départements n'est pas près de s'essouffler. ma question est simple : allez-vous écouter les propositions formulées par la profession agricole, qui demande à revoir la liste des critères de zonage, notamment paysagers, et permettre ainsi une répartition plus juste de cette cartographie ? La parole

Il faut aussi tenir compte des contraintes réglementaires et budgétaires à l'échelon européen, qui font qu'il n'y a aucune part d'arbitraire possible pour intégrer ou exclure tel ou tel territoire, pas plus qu'il n'y en a aujourd'hui pour repousser les échéances. Des discussions ont été engagées depuis 2016 avec les professionnels agricoles et les régions, afin d'établir ce nouveau zonage. À l'heure où je vous parle, madame la sénatrice, ces discussions se poursuivent avec l'appui de l'ensemble des services du ministère. Le zonage envisagé à l'issue d'un premier cycle de travail

et certains critères retenus n'étaient pas justifiables à l'échelon européen. Je recevrai demain les représentants professionnels de votre région pour faire le point sur cette situation. Nous héritons d'un dossier ancien. Nous avons fait le tour du sujet sur le plan technique, il nous faut maintenant sortir. L'objectif du Gouvernement est de parvenir à une cartographie à la mi-février, comme l'a demandé le Président de la République. Nous veillerons à la partager et à définir les mesures d'accompagnement, puis nous la transmettrons à la Commission européenne pour

Ils constituent un élément fort pour notre territoire et nous devons les accompagner. Actuellement, alors que les GAFA sont en train de piller le commerce, sans aucune contrepartie d'aucune sorte, taxe foncière, taxe d'habitation ou taxe sur la valeur ajoutée- rien, pas d'impôt

les encours et les prêts qu'elles ont consentis aux entreprises pour leur développement ont augmenté de plus de 5 %, ce qui est aussi le signe d'un retour de la croissance. Enfin, vous avez interrogé le Gouvernement sur la façon dont la taxe d'habitation sera compensée pour les collectivités. Engagement a été pris, et il sera tenu,

protestent contre la future carte des zones défavorisées simples que vous allez présenter prochainement à l'échelon européen. Or, en l'état, ce nouveau zonage, établi à partir de critères modifiés, exclura un grand nombre de communes jusqu'alors éligibles à ces aides européennes, qui étaient perçues par ces agriculteurs pour compenser le handicap naturel

la fin de ce type d'exploitation et, plus généralement aussi, la fin d'un certain type d'activités, dans ces zones si difficiles, où des paysans contribuent depuis si longtemps au maintien de nos paysages et à la vie de nos petites communes. Monsieur le ministre, quelles garanties et quels engagements fermes et tangibles pouvez-vous apporter aujourd'hui en ce qui concerne le maintien de ces aides vitales à nos agriculteurs ?

Je le répète, je recevrai des représentants demain pour faire un point précis de la situation avec eux. Nous étudierons les mesures d'accompagnement à mettre en place dans le souci de l'efficacité de nos politiques publiques. Nous devons collectivement nous tourner vers l'avenir. Monsieur le

La séance est reprise. J'ai le regret de vous faire part du décès de notre ancien collègue Claude Prouvoyeur, qui fut sénateur du Nord de 1983 à 1992. groupe socialiste et républicain, de la proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, présentée par Mme Nicole Bonnefoy et les membres du groupe socialiste et républicain

madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, en 2012, j'ai eu l'honneur d'être nommée rapporteur de la mission commune d'information sénatoriale sur les pesticides et leurs conséquences sur la santé

des conséquences de l'utilisation massive des pesticides dans notre pays. Chose suffisamment rare pour être soulignée, ce rapport fut alors adopté par le Sénat à l'unanimité. Depuis, un nombre important de recommandations ont été traduites dans la loi, parmi lesquelles l'instauration d'un suivi des produits pesticides après leur mise sur le marché ; l'interdiction de l'utilisation des pesticides dans les collectivités ; l'interdiction de leur vente aux particuliers en place du dispositif de phytopharmacovigilance, lequel permet d'instaurer une veille sanitaire dans tout le pays et de faire progresser l'évaluation des risques, des maladies et des produits mis sur le marché ; l'introduction dans notre droit de l'action de groupe en matière environnementale

contribué à tous ces progrès. En parallèle, la problématique des pesticides n'a cessé d'être confirmée et amplifiée. Outre la prise de conscience sociétale qui n'a fait que croître, je pense en particulier à la publication de plusieurs rapports ayant

liés à des expositions pour de nombreuses pathologies graves : plusieurs cancers- du sang, de la prostate, du cerveau, de la peau -, des troubles cognitifs et des maladies neurologiques- Parkinson, Alzheimer ... -, des maladies respiratoires et des troubles de la reproduction et du développement. Enfin, l'étude insiste fortement sur les risques pour le développement de l'enfant liés aux expositions au cours de la petite enfance et des périodes prénatale et périnatale. Deuxième rapport : celui de l'ANSES, notre agence nationale de sécurité sanitaire. Elle s'est penchée en 2016 sur les expositions professionnelles aux pesticides en agriculture. Alors que la consommation de pesticides est en progression constante, l'agence souligne que les données sur l'exposition aux pesticides sont « fragmentées » et « lacunaires ». Cette absence de transparence produit une « invisibilité des problèmes », un « relatif silence » sur les maladies professionnelles. Celui-ci s'explique entre autres éléments par les obstacles que rencontrent les malades qui souhaitent faire reconnaître leurs pathologies chroniques. L'ANSES ajoute que les éléments fournis par les industriels avant la mise sur le marché d'un pesticide ne suffisent pas mesurer son degré de dangerosité. Les études ne sont en effet pas publiées dans des revues scientifiques. Elles ne reposent ni sur des statistiques agricoles, ni sur des enquêtes de terrain, ni sur les déclarations individuelles. Elles ne reflètent pas l'éventail des situations réelles. Enfin, le dernier rapport en date sur ces questions a été publié en décembre 2017. Il achève de dresser un panorama éloquent de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans notre pays. Il s'agit du rapport des trois inspections générales des ministères de l'environnement, de la santé et de l'agriculture commandé par ce gouvernement. les points suivants : l'ensemble des citoyens sont potentiellement exposés aux pesticides, la quasi-totalité des cours d'eau sont contaminés, de nombreuses substances parmi les plus nocives sont encore autorisées à la vente en raison des impérities du dispositif européen d'autorisation,

L'inspection générale appelle à augmenter significativement l'effort financier en matière de recherche et à bâtir « un plan d'action visant à une sortie la plus rapide des produits phytos puisque « l'objectif d'une diminution rapide de leur utilisation constitue désormais un impératif pour la protection de la population ». C'est donc en toute logique que nous attendons du Gouvernement qu'il agisse conformément aux recommandations de ces divers rapports. Je suis, madame la ministre, d'autant plus optimiste que j'ai en mémoire les propos tenus le 12 juillet 2017 par Nicolas Hulot venu présenter au Sénat les « objectifs du développement durable » de son gouvernement. Il a alors que la santé environnementale était une priorité gouvernementale. « J'ai à coeur, a-t-il dit, de protéger la santé des agriculteurs contre l'utilisation abusive d'intrants. Je connais suffisamment d'agriculteurs victimes de pathologies lourdes qui sont abandonnés par ceux qui sont censés les soutenir. » Je ne doute pas que Nicolas Hulot pensait alors en particulier au soutien de l'État et du Gouvernement. Le texte que nous examinons aujourd'hui vise en premier lieu à protéger et à défendre les malades des pesticides, au premier rang desquels, j'y insiste, les agriculteurs. Trop souvent montrés du doigt pour l'utilisation de ces produits, ils sont les premiers et les plus nombreux à souffrir de leurs effets nocifs. Les maladies liées aux expositions aux pesticides font l'objet d'un phénomène massif de sous-déclaration et, donc, de sous-reconnaissance. Dans son rapport de 2016, l'ANSES mettait en regard deux chiffres essentiels : d'une part, plus de 1 million de personnes sont professionnellement exposées en France aux pesticides ; d'autre part, entre 2002 et 2010, seulement 47 maladies professionnelles de ce type ont en tout et pour tout été reconnues.

Je tiens ici à les saluer, ainsi que leur président, Paul François, et l'avocat M Lafforgue, qui ont très largement contribué à l'écriture de ce texte. Paul François a été intoxiqué en 2004. Or le lien entre ses troubles et son exposition n'a été reconnu qu'en 2010.

Près de quinze ans après son empoisonnement aigu, son état de santé s'est dégradé. Aucuns dommages et intérêts ne lui ont été versés et son parcours judiciaire va encore durer plusieurs années. Est-ce juste, madame la ministre ?

Après plus de sept ans de procédures judiciaires pour faire reconnaître leur maladie professionnelle, plusieurs d'entre eux n'ont toujours rien obtenu, alors qu'ils ont, pour certains, perdu leur travail et sont arrivés au bout de leurs droits aux indemnités chômage. Ce qui est important, c'est que nous soyons reconnus. De toute façon, notre vie est gâchée. » Tels sont les terribles mots d'un ex-salarié, Claude Le Guyader, qui était encore avant-hier devant la cour d'appel du tribunal des affaires sociales de Rennes pour obtenir cette reconnaissance aux côtés de son collègue Pascal Brigand. Est-ce juste, madame la ministre ? Je pense encore aux innombrables victimes des épandages massifs de chlordécone et de paraquat, mon collègue Victorin Lurel parlera mieux que moi. Il est indispensable d'apporter une réponse juste aux terribles séquelles qui continuent d'affecter la Guadeloupe et la Martinique, à la suite des contaminations à ces substances, leur rémanence dans l'environnement étant de l'ordre de 600 ans et elles sont transmissibles de génération en génération. Est-ce juste, madame la ministre ? Le texte en discussion aujourd'hui a dès lors vocation à faciliter le parcours de reconnaissance et d'indemnisation de ces malades

madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, permettez-moi de commencer cette intervention par un double constat, dressé conjointement par trois corps d'inspection de l'État, dans un rapport rendu public le 19 janvier dernier. Je pense que nous pouvons tous ici le partager. souligne tout d'abord que l'utilisation massive des pesticides constitue « un enjeu majeur de santé publique tant pour les applicateurs et leurs familles que pour les riverains et la population en général ». Ce constat n'est pas nouveau. La mission d'information menée en 2012, présidée par notre collègue Sophie Primas et dont la rapporteur était Nicole Bonnefoy, faisait déjà état d'une « urgence sanitaire » sous-évaluée, notamment au regard des données épidémiologiques. Le rapport souligne en outre que « le degré de certitude d'ores et déjà acquis sur les effets des produits phytopharmaceutiques commande de prendre des mesures fortes et rapides, sauf à engager la responsabilité des pouvoirs publics ». Le message est clair. Les études scientifiques soulignent en effet que l'exposition des travailleurs et de leurs familles à ces produits augmente de manière significative les risques de contracter certaines pathologies. En France, l'expertise collective de l'INSERM de 2013, fondée sur une revue de la littérature scientifique internationale publiée au cours des trente dernières années, met au jour plusieurs niveaux de présomption s'agissant du lien entre l'exposition aux pesticides et différentes pathologies : hémopathies malignes, tumeurs cérébrales, cancers cutanés, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs ou encore certains troubles de la reproduction et du développement. Elle insiste par ailleurs sur les expositions au cours de la période prénatale et périnatale, ainsi que pendant la petite enfance, qui semblent être particulièrement à risques pour le développement de l'enfant. Nous savons que, sur certains points fondamentaux, les connaissances scientifiques établies permettent de retenir un lien de causalité : au sein du régime agricole, les quinze tableaux de maladies professionnelles liées à l'exposition aux pesticides sont là pour nous le rappeler. La proposition de loi déposée par notre collègue Nicole Bonnefoy s'inscrit dans le prolongement de ces constats et pose la question de la réparation des dommages. Elle prévoit, sous certaines conditions, l'indemnisation des préjudices résultant de l'exposition à des produits phytopharmaceutiques en allant au-delà de la simple réparation forfaitaire, que notre législation sociale limite aux victimes professionnelles. Les professionnels du secteur agricole sont bien évidemment la première population concernée.

pourront accéder au dispositif d'indemnisation dès lors qu'ils auront préalablement obtenu la reconnaissance d'une pathologie d'origine professionnelle sur le fondement du système déjà existant des tableaux de maladies professionnelles. Au regard des dommages causés, qui dépassent largement le préjudice économique pour englober les préjudices extrapatrimoniaux, une telle avancée me paraît aller dans le sens de l'histoire de notre protection sociale. Il en va de même de l'ouverture du dispositif aux victimes exposées en dehors du cadre professionnel et que l'on peut qualifier de « victimes environnementales ». Je pense notamment aux riverains de champs agricoles qui subissent les effets des épandages. La proposition de loi les inclut dans le dispositif. Elle couvre enfin les enfants atteints d'une pathologie occasionnée par l'exposition aux pesticides de l'un de leurs parents. Il s'agit ici de prendre en compte principalement les expositions. De De manière générale, il est apparu au cours des auditions que j'ai menées que la volonté d'améliorer les règles d'indemnisation est accueillie très positivement. L'ANSES, en particulier, s'est montrée favorable à la recherche d'une plus grande équité dans la prise en charge des victimes. pourquoi les victimes de l'amiante, des irradiations dues aux essais nucléaires, de médicaments auraient-elles accès à une réparation intégrale alors que les agriculteurs victimes de produits phytopharmaceutiques sont limités à une réparation forfaitaire ? L'ANSES a également souligné l'avantage d'un tel dispositif, qui permet de limiter les inconvénients liés à une judiciarisation des demandes. Les réserves formulées sur la proposition de loi dans sa rédaction initiale ont essentiellement porté sur deux points la gouvernance du fonds d'indemnisation et la procédure d'instruction, qu'il a donc fallu préciser ; d'autre part, le financement, sur lequel les avis sont partagés. D'aucuns souhaiteraient que le financement soit entièrement étatique et craignent qu'une hausse de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques ne soit répercutée sur le prix de vente. Compte tenu du chiffre d'affaires du secteur en France- plus de 2 milliards d'euros chaque année -et de la capacité de négociation des intermédiaires, il me semble que cette réserve peut être levée. J'ajoute que les règles de recevabilité financière auxquelles nous sommes soumis ne nous permettraient pas de prévoir une contribution de l'État au financement du fonds. Une telle initiative, madame la ministre, ne pourrait venir que du Gouvernement. Si la fiscalité déjà prélevée sur la vente des produits phytopharmaceutiques offre un montant d'amorçage raisonnable, les ressources du fonds, nous en convenons tous, devront nécessairement être revues. La commission des affaires sociales a apporté plusieurs séries de précisions à la proposition de loi afin de parvenir à un encadrement juridique rigoureux, prudentiel et qui sera nécessairement appelé à évoluer. L'article 1 définit le champ des personnes éligibles au dispositif d'indemnisation. Sa rédaction initiale ne permettait pas d'en cerner parfaitement les contours. C'est pourquoi la commission a renvoyé à un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'agriculture le soin d'établir la liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation pour les victimes non professionnelles. À l'article 2, la commission a précisé l'organisation du fonds d'indemnisation en prévoyant qu'il comprend un conseil de gestion dont la composition est fixée par décret et qu'il est représenté à l'égard des tiers par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. agricole. Sur la procédure d'examen des demandes, la commission a partagé l'avis général selon lequel faire reposer la charge de la preuve sur le demandeur rendrait le dispositif extrêmement complexe et, pour tout dire, très difficilement accessible. La jurisprudence récente dans le domaine de la santé reconnaît aujourd'hui que le doute scientifique ne fait pas nécessairement obstacle à la preuve requise du demandeur dès lors que celui-ci fait valoir un faisceau d'indices concordants sur les dommages causés par le produit. Nous avons donc jugé préférable de retenir une présomption de causalité. Une commission médicale indépendante serait chargée d'examiner les circonstances des expositions et de statuer sur leur lien avec la pathologie. C'est d'ailleurs le modèle des dispositions en vigueur pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA. À l'article 4, la commission a porté de six à neuf mois le délai au terme duquel le fonds est tenu de présenter une offre d'indemnisation au demandeur. au demandeur. L'article 7, qui prévoyait que le fonds serait financé notamment par une fraction de la taxe sur la vente de produits phytopharmaceutiques, dispose désormais que le produit de cette taxe sera affecté en priorité à l'ANSES et, pour le solde, au fonds d'indemnisation. Aujourd'hui, la taxe sur les produits phytopharmaceutiques, collectée par l'ANSES, permet de financer le dispositif de phytopharmacovigilance. Il est essentiel que celui-ci soit totalement préservé. Enfin, au travers de l'article 9, la commission a renvoyé à un décret en Conseil d'État le soin de définir les modalités d'application de la loi et prévu une période transitoire durant laquelle le délai laissé au fonds pour présenter une offre est porté à douze mois au lieu de neuf. Il s'agit, sur ce point, de tenir compte des nécessaires contraintes liées à la phase d'installation et de montée en charge du fonds. président, madame la ministre, mes chers collègues, les principales modifications apportées par la commission à la proposition de loi initiale. Au cours de nos débats, je ne doute pas que certains souhaiteront insister sur l'encadrement plus étroit dont les produits phytopharmaceutiques ont progressivement ont progressivement fait l'objet au cours des dernières décennies. Je rappellerai simplement à ce stade que la nécessité de renforcer la prévention et la protection,

pour ne pas différer notre travail de législateur au motif que ces connaissances sont encore en progrès. Il y va de notre responsabilité commune. La parole

nous le savons, les scandales sanitaires sont au nombre des menaces qui pèsent le plus lourdement sur notre démocratie, tant ils entament la confiance des Français. Votre proposition de loi vise à répondre à un impératif de santé publique et de reconnaissance du préjudice subi. Vous souhaitez créer un fonds assurant la réparation intégrale des victimes de pathologies liées aux produits phytopharmaceutiques, que leur exposition soit d'origine professionnelle ou environnementale. Ce fonds serait financé exclusivement par une taxe prélevée sur les produits concernés. Votre texte, mesdames, messieurs les sénateurs, est empreint d'une noble intention, et je la comprends. Toutefois, la création d'un tel fonds d'indemnisation m'apparaît prématurée. En effet, nous connaissons encore trop mal les risques sur la santé d'une exposition à un ou plusieurs produits phytopharmaceutiques. Les pathologies en question, vous le savez, peuvent avoir plusieurs causes. Aussi ne peuvent-elles être directement imputées, en tous les cas pour la majorité d'entre elles, aux seuls produits phytopharmaceutiques. Ce dispositif renverserait la charge de la preuve. Ce serait alors au fonds de démontrer l'absence de lien direct et essentiel entre une pathologie et les expositions, dès lors que la victime alléguerait une exposition. Or, compte tenu de l'utilisation massive des pesticides, il convient de considérer que tout le monde est exposé : le champ des indemnisations s'étendrait aux victimes environnementales, et ce de façon difficilement contrôlable. Par ailleurs, un tel dispositif d'indemnisation serait, à mes yeux, déresponsabilisant, en particulier vis-à-vis des industriels. Les effets sur la santé des expositions professionnelles aux produits phytopharmaceutiques font l'objet d'un consensus scientifique. Or votre texte s'engage sur la voie d'une indemnisation systématique, sans détermination préalable de responsabilité. En outre, cette indemnisation serait financée exclusivement par le produit d'une taxe sur les produits phytopharmaceutiques. Malgré l'intention qui vous anime, les industriels bénéficieraient, de fait, d'une décharge de responsabilité individuelle contre une prise en charge mutualisée du risque. Nous devons plutôt renforcer l'indemnisation dans le cadre du système des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ce système facilite l'indemnisation des victimes concernées. En effet, lorsqu'une maladie est inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et répond aux conditions prévues par ce tableau, elle est présumée d'origine professionnelle. Qui plus est, pour les maladies n'étant pas inscrites dans les tableaux, une voie complémentaire de reconnaissance permet un examen, au cas par cas, des demandes par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, les CRRMP. Au total, pas moins de 700 maladies professionnelles, liées aux produits phytopharmaceutiques, sont reconnues dans ce cadre. Cela étant, je suis évidemment consciente des limites de ce système d'indemnisation. En effet, comme vous le dites très justement, il ne permet pas à tous les travailleurs concernés d'être indemnisés de manière équitable. Les tableaux de maladies professionnelles existants n'ont pas été actualisés au regard des connaissances scientifiques les plus récentes. Je pense en particulier à l'expertise collective de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale- INSERM -de 2013. Quant aux maladies non inscrites dans les tableaux, les décisions rendues après avis des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles sont hétérogènes, les connaissances scientifiques n'étant pas assez diffusées. Afin de résoudre ces écueils, Mme la ministre du travail, M. le ministre de l'agriculture et moi-même demanderons aux commissions chargées d'élaborer ces tableaux d'améliorer l'indemnisation des travailleurs concernés. Précisément, des études devront être menées pour adapter les tableaux de maladies professionnelles à l'état actuel des connaissances scientifiques. Toutefois, au-delà de l'indemnisation elle-même, la priorité ira à la prévention des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé. La feuille de route du Gouvernement, à la suite du rapport sur les produits phytosanitaires, doit renforcer l'effort de recherche afin de mieux connaître les liens entre pathologies et exposition, mais également de développer les actions de protection des travailleurs et des et des populations. Je pense en particulier aux publics les plus fragiles et les plus vulnérables, les enfants et les femmes enceintes. Nous devons également étudier les conclusions du rapport de la mission diligentée auprès de l'inspection générale des affaires sociales, de l'inspection générale des finances et du conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, rapport qui vient de m'être communiqué et qui étudie l'éventualité d'un dispositif d'indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques. Nous avons besoin de temps pour analyser les conclusions de ce rapport, ainsi que les enjeux juridiques, financiers et sociaux de ses propositions. Cela étant, ce rapport semble pointer l'absence de certitudes scientifiques sur le lien de causalité entre maladie et exposition à des substances nocives, ce qui, comme je le disais, constitue le principal obstacle à la reconnaissance des victimes environnementales. Le rapport Devant cette difficulté de démonstration du lien de causalité pour un nombre de victimes important, l'amélioration du régime accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP) par extension du périmètre des maladies prises en charge, pour le rendre cohérent avec l'évolution des connaissances scientifiques, pourrait être une option possible. Par ailleurs, le plan santé au travail 3, élaboré par les partenaires sociaux, prévoit des actions de substitution de certains produits phytopharmaceutiques, ainsi qu'un travail sur le port d'équipements de protection pour les travailleurs. Quant aux amendements visant à intégrer la problématique du chlordécone aux Antilles, je crains qu'ils n'engendrent une confusion avec le plan Écophyto ... C'est un échec ! ... et les études épidémiologiques en cours de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et de Santé publique France.

Si nous incluons dans le dispositif un lien entre utilisation des produits phytopharmaceutiques et une pollution, et non plus un lien entre une exposition et une indemnisation, nous ferons perdre au fonds sa vocation essentielle d'indemniser des personnes. Soyez assurés, mesdames, messieurs les sénateurs, que mon ministère fera face à cet enjeu, fort des conclusions du comité de pilotage de décembre dernier. J'attends également de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, qu'elle précise la position qu'elle a rendue, à la suite de son rapport du 15 décembre dernier. Pour autant, c'est au plan chlordécone de traiter les questions relatives au chlordécone. J'ai toute confiance dans les vertus de ce plan, dont le principal mérite est de passer d'une logique de gestion de court terme des effets collatéraux de la pollution à une véritable logique de long terme de développement durable des territoires, intégrant la problématique du chlordécone. L'inspection générale de l'administration souligne elle-même l'efficacité du dispositif : sa grande souplesse permet de réagir avec diligence pour répondre aux besoins de terrain. En tout état de cause, je m'attacherai à ce que mes services répondent sur le fond et très précisément à l'ensemble des questions techniques qui m'ont été posées sur le risque chlordécone, dont certaines ont été fort justement relayées par des parlementaires. Mesdames, messieurs les sénateurs, l'actualité des enjeux liés aux produits phytosanitaires exige de nous de la résolution, mais aussi de la préparation. À la remise du rapport inter-inspections doit dorénavant succéder une analyse interministérielle de fond, animée par la patience de la réflexion. Par ailleurs, la concertation sur une feuille de route relative à ces sujets vient tout juste d'être lancée : laissons-lui le temps de mettre en place les actions qui conviennent. Les Français exigent certes de la résolution, mais aussi de la lisibilité. C'est pourquoi les travaux à venir doivent s'inscrire dans un cadre déjà défini, celui de la feuille de route sur les produits phytosanitaires et du plan Écophyto. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui autour d'un sujet de première importance : la protection de la santé des Français face à la dangerosité de certains produits phytopharmaceutiques. En 2012, une mission sénatoriale, présidée par notre collègue Sophie Primas et dont vous avez été, madame Bonnefoy, la rapporteur, avait alerté notre hémicycle sur l'urgence de ces sujets et proposé une centaine de recommandations pour lutter contre les pesticides cancérigènes.

La question dépasse en effet les clivages partisans. Après sept mois d'auditions, la mission avait conclu à une sous-évaluation des dangers relatifs aux pesticides, à une insuffisante prise en compte du suivi des produits après leur mise sur le marché et à un manque de prise en compte des problématiques de santé dans les pratiques industrielles, agricoles et commerciales actuelles. Ce rapport avait été un véritable signal d'alarme pour le précédent gouvernement : l'Institut national de la santé et de la recherche médicale s'était saisi du sujet, publiant lui-même un rapport en juin 2013, et la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt d'octobre 2014 avait mis en place un dispositif de phytopharmacovigilance. Cette loi avait aussi marqué un tournant important de notre approche de ce sujet, en reconnaissant les hémopathies en lien avec l'exposition professionnelle aux pesticides comme des maladies professionnelles. la présente proposition de loi entendent aller plus loin. En complétant ce dispositif avec une prise en charge de la réparation intégrale des préjudices des personnes atteintes de maladies liées à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, ils souhaitent que soient reconnus les dangers de ces produits et la réalité de ces pathologies. Comme cela fut le cas en leur temps pour les victimes de l'amiante ou les vétérans des essais nucléaires, la création d'un fonds d'indemnisation permettra de reconnaître la réalité de la maladie et de sensibiliser la population à ce problème récurrent. Aujourd'hui encore, devant les tribunaux, de nombreux salariés agricoles plaident pour faire reconnaître leurs pathologies comme des maladies professionnelles. Il faut à mon avis les accompagner dans ce combat de tous les jours. de deux ex-salariés de la coopérative agricole Nutréa-Triskalia, atteints d'hypersensibilité aux produits chimiques à la suite de leur surexposition, déclarés inaptes au travail et finalement congédiés. En septembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Brieuc avait jugé la coopérative coupable d'une faute inexcusable pour l'intoxication de ses employés en 2010. La décision avait fait grand bruit. En décembre 2017, encore, le conseil des prud'hommes de Lorient a déclaré leur licenciement sans cause réelle et sérieuse. En réaction, le commissaire européen chargé de la santé et de la sécurité alimentaire, Vytenis Andriukaitis, a demandé la tenue d'un audit sur les pratiques des entreprises agroalimentaires bretonnes au printemps 2018. de la proposition de loi, mes chers collègues, devrait nous permettre de répondre à ce genre de situation. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le groupe Les Indépendants attire votre attention sur l'importance de cette proposition de loi dans la reconnaissance de l'un des fléaux modernes du monde agricole : la dangerosité des produits utilisés. Elle recueille son soutien. Elle répond à une inquiétude de terrain, dont de nombreux agriculteurs ont fait la désagréable expérience, et elle a, jusqu'à présent, fait l'objet d'une relative unanimité dans nos débats.

J'en retiendrai trois. En premier lieu, vous évoquez l'incertitude qui pèse sur le lien de causalité actuel de telle ou telle molécule. Je comprends le problème de la charge de la preuve qui peut s'y attacher.

du constat est différé. On peut compter, je dois le dire, sur les industriels et sur les lobbies pour faire en sorte que les preuves de toxicité

pas été inutile. Il aura constitué une étape de plus dans la lutte contre le scandale de l'exposition aux pesticides, au côté duquel celui du Mediator ou du Vioxx risque d'apparaître, demain, une fois que la lumière sera faite entièrement,

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, utilisés pour protéger les cultures, limiter la propagation de parasites et améliorer la qualité de la production alimentaire, les pesticides sont au coeur du développement agricole des cinquante dernières années. comme le rappelle notre collègue Nicole Bonnefoy dans son rapport, « Le formidable succès des pesticides et la banalisation progressive de leur emploi ne doit pas faire perdre de vue leur raison même d'exister : les pesticides sont conçus pour tuer. Les rapports dénonçant les dangers des produits phytosanitaires sur l'environnement et la biodiversité sont bien connus. La France, premier pays européen et troisième mondial pour l'utilisation de pesticides, a engagé des mesures de prévention dans ce domaine, notamment avec la mise en place, en 2014, d'un système de pharmacovigilance. C'est une bonne chose. Mais cela ne règle pas la question des personnes déjà malades, ni de celles qui le seront demain. Car les rapports scientifiques montrant les liens entre certaines pathologies et l'exposition aux pesticides se multiplient également. Nous avons aujourd'hui la certitude que ces produits, une contamination par l'air, l'eau, le sol et l'alimentation, ont des effets sur le développement du foetus, de maladies aiguës et chroniques, ou encore sur le développement neurologique. Lors d'une audition à l'Assemblée nationale en novembre 2017, la mutualité sociale agricole ont reconnu que 2 % des maladies professionnelles des agriculteurs étaient liées à des produits phytosanitaires. En 2016, 61 assurés se sont vu reconnaître une maladie professionnelle provoquée par l'utilisation de pesticides 25 hémopathies malignes et 36 maladies de Parkinson. Il s'agit bien d'un enjeu sanitaire majeur. Comme l'a rappelé l'auteur de la proposition de loi, ce texte « vise en premier lieu à protéger et défendre les malades des pesticides, au premier rang desquels les agriculteurs, trop souvent montrés du doigt pour l'utilisation de produits dont ils sont les plus nombreux à souffrir des effets nocifs deux pathologies sont actuellement inscrites dans le tableau des maladies professionnelles agricoles, les associations ne dénombrent pas moins de 180 cas de pathologies déclarées dues à ces produits. Les agriculteurs ne sont toutefois pas les seules victimes des pesticides. Les familles et les riverains sont également exposés. Bien qu'un arrêté de 2006 oblige les agriculteurs à mettre en oeuvre les moyens appropriés pour éviter que les produits phytopharmaceutiques ne soient entraînés en dehors de la parcelle ou de la zone traitée, force est de constater que les riverains d'exploitations agricoles sont aussi en première ligne. Aujourd'hui, 14 millions de Français vivent en zone rurale et nombre d'entre eux à proximité immédiate de ces exploitations. Si l'ampleur réelle de leur exposition aux produits phytosanitaires est encore méconnue, l'INSERM, dans le cadre d'une expertise collective menée en 2013, évoque une augmentation du risque de malformations congénitales, de tumeurs cérébrales et de leucémies chez les enfants des femmes vivant au voisinage d'une zone agricole. Le Gouvernement vient de présenter un projet de plan d'action pour interdire le plus rapidement possible les substances les plus préoccupantes et réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques. Il faudra également que la France puisse faire évoluer le droit européen pour inciter chaque État à retirer ces substances dès que des alternatives seront trouvées. Dans cette attente, les victimes ne peuvent plus être ignorées : nous devons leur proposer des mesures d'accompagnement et d'indemnisation, une meilleure reconnaissance des conséquences, sur la santé, de produits jusqu'à présent autorisés par l'État. Comme l'a très justement exprimé le rapporteur, Bernard Jomier : « [La] nécessité de renforcer la prévention, dont chacun partage le constat, n'épuise pas le sujet de la réparation lorsque des dommages ont été subis. Européen, sensible à ces arguments et favorable à la création d'un fonds d'indemnisation, votera donc en faveur de cette proposition de loi. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques constitue aujourd'hui un enjeu majeur de santé publique. En effet, il ressort de différentes études publiées ces dernières années des augmentations de risques significatives pour plusieurs pathologies, en lien avec l'exposition des travailleurs et de leurs familles. Le Sénat s'est saisi, dès 2012, de cette problématique et a créé une mission d'information, présidée par Sophie Primas et rapportée par Nicole Bonnefoy. La mission a dressé plusieurs constats les dangers et les risques des pesticides pour la santé sont sous-évalués ; le suivi des produits après leur mise sur le marché n'est qu'imparfaitement assuré au regard de leurs impacts sanitaires réels ; les protections contre les pesticides ne sont pas à la hauteur des dangers et des risques ou encore, le fait, mais c'était il y a plus de cinq ans, que les pratiques industrielles, agricoles et commerciales n'intègrent pas suffisamment ces préoccupations. Actuellement, notre législation rend possible l'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques en cas de reconnaissance d'une maladie contractée dans le cadre professionnel. Les exploitants et les salariés agricoles disposent de tableaux de maladies professionnelles spécifiques au régime agricole. Une dizaine de tableaux concernent l'exposition aux produits phytosanitaires. L'ensemble du système repose sur une présomption d'imputabilité pour les personnes ayant travaillé au contact de certains risques répertoriés et constatant l'apparition d'une pathologie dans un délai déterminé. Cependant, il est vrai que le dispositif de réparation paraît aujourd'hui insuffisant et inéquitable. Partant de ce constat, la proposition de loi dont nous débattons cet après-midi instaure un dispositif de réparation intégrale. Pour ce faire, ses auteurs proposent la création d'un fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques. Le texte prévoit que ce fonds soit géré par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et financé par l'attribution d'une fraction de la taxe prévue à l'article L. Je rappelle que la loi de finances rectificative pour 2014 a en effet introduit une nouvelle taxe sur les produits phytopharmaceutiques perçue au profit de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, afin de financer le dispositif de phytopharmacovigilance, qui vise à identifier les effets indésirables des produits phytopharmaceutiques. Un arrêté du 27 mars 2015 fixant le taux de la taxe sur les ventes de produits phytopharmaceutiques a prévu un taux à 0,2 % du chiffre d'affaires, réduit à 0,1 % pour les produits de biocontrôle. Cependant, et c'est mon premier point, je m'interroge sur ce financement, qui me semble bien insuffisant. Monsieur le rapporteur, vous avez évoqué un besoin de 10 millions d'euros pour financer ce fonds. La taxe actuellement affectée à l'ANSES rapporte 4 millions d'euros par an. Une fraction de cette taxe ne peut suffire à financer le dispositif. Par ailleurs, la MSA a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas gérer ce fonds, pas plus que la CNAM. Sans oublier que les syndicats agricoles craignent qu'une hausse de la taxe ne soit répercutée sur le prix de vente. Deuxième point, le texte définit un champ des personnes éligibles au dispositif d'indemnisation plutôt large

Certes, monsieur le rapporteur, la commission a adopté un amendement qui visait à renvoyer à un arrêté ministériel le soin d'établir la liste des pathologies ouvrant droit à indemnisation pour les victimes non professionnelles. Mais le champ reste large. Comment estimer le nombre de victimes potentiellement concernées ? Troisième point, enfin, le texte dispose que le demandeur justifie d'un lien direct entre son exposition aux pesticides et la pathologie. Monsieur le rapporteur, vous avez proposé de transformer la charge de la preuve reposant sur le demandeur en présomption de causalité et souhaitez renvoyer à une commission médicale indépendante la mission d'examiner les circonstances des expositions et de statuer sur leur lien avec la pathologie. Il s'agit d'un dispositif qui s'inspirerait des dispositions en vigueur pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, le FIVA. cette comparaison avec le FIVA est intéressante, elle ne peut être totale. Le lien entre amiante et pathologie- plaques pleurales ou mésothéliome -est facile à établir. Je rappellerai que le FIVA est financé par la branche AT-MP, donc par les entreprises, et que le financement par l'État est réduit chaque

2017. Elle recommande d'actionner nombre de leviers, que je ne vais pas détailler, pour réduire de façon pérenne la dépendance aux produits phytopharmaceutiques. Le modèle de production agricole qui s'est développé après-guerre reposait en effet sur cette dépendance. Nos exploitants agricoles ont pris conscience des dangers liés à l'utilisation de ces produits et s'acheminent vers leur moindre utilisation. Nous devons les accompagner dans cette démarche. Les entreprises du secteur des produits phytosanitaires orientent leurs recherches en vue de changer les molécules. La recherche agronomique se mobilise pour trouver des alternatives. La MSA s'investit dans la prévention, la formation et entame une évolution du tableau des maladies professionnelles. Cette proposition de loi, comme l'a dit notre collègue Claude Malhuret, permet d'appeler le débat au Sénat sur un sujet majeur. J'en remercie l'auteur et le rapporteur. Bien entendu, la question de l'indemnisation se pose et doit trouver un mode de réparation adapté. Néanmoins, pour les raisons que je viens d'évoquer, notre groupe, dans sa grande majorité, s'abstiendra.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les effets sur la santé de l'exposition aux pesticides suscitent de fortes et légitimes inquiétudes dans l'opinion. Cette question de santé publique est inscrite depuis plusieurs années à l'agenda politique national et européen. Ainsi, le rapport d'information de notre collègue Nicole Bonnefoy a permis de formuler des recommandations pour renforcer la sécurité de l'utilisation de ces produits et les connaissances de leurs effets. le plan européen, l'actualité récente a mis sur le devant de la scène la question de l'interdiction des perturbateurs endocriniens et la reconduction de l'autorisation du glyphosate. À cet égard, je me permets de vous signaler les travaux de la commission des affaires européennes de notre assemblée, que j'ai eu l'honneur de conduire avec notre ancien collègue Alain Vasselle. Les risques sont encore plus forts chez les exploitants agricoles et tous les professionnels amenés à manipuler, parfois massivement, de nombreuses substances tout au long de leur carrière. Dans un rapport de 2016, l'ANSES a rappelé l'ampleur de la population concernée : « En 2010, plus d'un million de personnes avaient une activité régulière en agriculture, auxquelles doivent être ajoutées plusieurs centaines de milliers de travailleurs non permanents, ainsi que plusieurs dizaines de milliers de stagiaires.

utile, la densité moyenne d'usage de pesticides en France à 2,9 kilogrammes de substance active à l'hectare, nous plaçant ainsi dans la moyenne européenne. Cette expertise collective de l'INSERM en 2013 a conclu que de nombreuses études épidémiologiques mettaient en évidence une association entre les expositions aux pesticides et certaines pathologies chroniques, notamment certains cancers, certaines maladies neurologiques et certains troubles de la reproduction et du développement. Selon les cas, les niveaux de présomption peuvent aller de faible à fort. Par ailleurs, des travaux de recherche ont attiré l'attention sur les effets éventuels d'une exposition, même à faible intensité, lors de périodes sensibles du développement, et pendant l'enfance. Devant de tels constats, nous sommes tous conscients qu'il faut appliquer avec la plus grande détermination des mesures de prévention, y compris par l'interdiction si nécessaire. Plus généralement, il nous il nous faut réduire dès maintenant la dépendance de notre agriculture aux produits phytosanitaires. Le Gouvernement agit concrètement en ce sens : le projet de loi Agriculture,

et de conseil en la matière, qui conduisent à une ambiguïté et des compensations entre les deux métiers. Si tout doit être fait pour éviter l'exposition aux pesticides, il faut déployer la même détermination s'agissant de la réparation des victimes. L'objectif de cette proposition de loi est de compléter le dispositif actuel de réparation, fondé sur la reconnaissance des maladies professionnelles. Il faut reconnaître que le système actuel n'est pas en mesure de répondre aux enjeux. On ne peut en effet se satisfaire du très faible taux de reconnaissance des maladies professionnelles liées aux pesticides, de la longueur des procédures induites, surtout lorsqu'elles s'accompagnent d'une phase judiciaire. Ajoutons que la réparation, quand elle est finalement obtenue, ne couvre pas le préjudice économique subi par les victimes. Le texte prévoit donc de créer un fonds d'indemnisation, alimenté par la taxe sur les produits phytosanitaires, qui assurerait une réparation intégrale du préjudice subi après l'avis d'une commission médicale. Le groupe La République En Marche s'associe à la volonté de l'auteur de la proposition de loi de rechercher plus de rapidité dans la procédure et plus de générosité dans l'indemnisation. Les amendements adoptés en commission ont permis de préciser des points importants du dispositif. Notre groupe s'était abstenu au stade de l'examen en commission, considérant qu'avant de créer un tel fonds il convenait de réformer le dispositif existant et d'améliorer et de compléter les tableaux de maladies professionnelles. Nous partageons les problématiques que soulève le texte aujourd'hui. C'est un texte d'appel, madame la ministre, pour qu'ensemble, avec le Gouvernement, les caisses concernées et les industriels, nous trouvions une solution durable et effective pour les victimes des pesticides. nous avons entendu vos arguments, qui tiennent compte de l'importance de ce dossier. Cette proposition de loi étant incomplète, en particulier dans le système d'indemnisation, notre groupe vous fait confiance pour trouver les solutions les plus adaptées aux victimes. C'est pourquoi, en l'état du texte, nous nous abstiendrons.

Les pesticides et leurs effets sur la santé sont devenus, à juste titre, un sujet de préoccupation pour nos concitoyennes et nos concitoyens, une véritable question de santé publique. Pendant des décennies, les fabricants de de produits phytosanitaires ont promis aux agriculteurs que l'emploi de ces produits leur permettrait d'obtenir des rendements des plus intéressants sans prise de risque particulière sur la santé. Pendant longtemps, rien n'indiquait, sur les bidons utilisés, la dangerosité des produits. Pendant longtemps, les agriculteurs ont versé à mains nues des pesticides dans leur cuve, ont déambulé en plein épandage sans masque ni combinaison. L'Union des industries de la protection des plantes, le lobby des fabricants de pesticides, renvoyait même les agriculteurs victimes aux précautions qu'il fallait prendre pour manipuler ces produits. Des dizaines d'études épidémiologiques menées sur toute la planète ont fait la démonstration que les utilisateurs de pesticides sont plus souvent atteints par certains cancers que la population générale. Je rappellerai que, d'après l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les expositions aux pesticides au cours de la période prénatale,, et périnatale, ainsi que pendant la petite enfance, présentent des risques pour le développement de l'enfant.

Les alternatives techniques aux pesticides existent. Pour sortir de l'utilisation en masse de ces produits phytosanitaires, il faut avant tout oser affronter la logique de compétition sur les prix à laquelle les paysans doivent faire face pour obtenir un revenu. d'une question écrite du 21 décembre dernier, ma collègue Christine Prunaud vous a interpellée, madame la ministre, concernant l'interdiction de l'utilisation de pesticides et d'insecticides dans les filières de l'agroalimentaire. En attendant cette interdiction, nous pensons que les victimes doivent être prises en charge. La proposition de loi de nos collègues socialistes et républicains s'insère dans la continuité de la création, en 2014, d'un système de pharmacovigilance. Elle prévoit de compléter ce dispositif en créant un fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides, comme cela a été fait pour les victimes de l'amiante ou des essais nucléaires. Elle va dans le sens d'une juste réparation des dommages des victimes au même titre que les maladies professionnelles. Il faut le rappeler, si les agriculteurs et les salariés agricoles sont les premières victimes de pesticides, l'exposition concerne aussi les salariés de l'agroalimentaire, ceux qui oeuvrent dans les usines de traitement du bois ou encore des milliers de travailleurs qui ouvrent au quotidien des conteneurs et y pénètrent pour des contrôles ou de la manutention. il paraît indispensable que l'exposition aux pesticides soit étendue au-delà des seuls professionnels, car, en réalité, l'ensemble des citoyens sont concernés à des degrés divers. C'est d'ailleurs ce que vous avez souligné, madame la ministre. Je pense bien sûr non seulement au voisinage des champs traités, mais également aux produits alimentaires que nous consommons. Il est en outre primordial que le fonds soit ouvert aux enfants malades du fait de l'exposition de leurs parents.

Et si le nombre de demandes est trop important, comme vous semblez le craindre, madame la ministre, il sera toujours temps de revoir la contribution des entreprises de produits phytopharmaceutiques en taxant leurs profits. En attendant, la réparation des préjudices liés à l'utilisation de ces produits s'inscrit dans la lutte pour la reconnaissance des nouvelles maladies professionnelles et leur indemnisation. Je ne partage pas votre prudence, madame la ministre. Bien sûr, chaque jour, les progrès des sciences nous permettent de nouvelles découvertes. Mais attendre est une prise de risques aux conséquences graves, voire mortelles. Ne laissons pas les lobbies des fabricants de pesticides continuer à répandre leur poison. D'autant que nous n'en sommes pas à l'année zéro, des avancées ont déjà été faites dans ce domaine. Vous avez ainsi mandaté un certain nombre de commissions de réflexion, c'est une bonne chose. Mais pourquoi ne pas prendre en compte la présente proposition de loi ?

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui nous concerne tous. Elle est des plus délicates à aborder, tant le sujet est douloureux pour bon nombre de nos concitoyens. Les produits phytopharmaceutiques sont utilisés pour favoriser la réalisation d'une agriculture intensive, qui ne permet plus aux agriculteurs de vivre dignement. Ces pratiques ont des conséquences sur la santé de ceux qui les manipulent et, au-delà, sur celle des riverains et sur l'environnement. Je ne parle pas des conséquences, en bout de chaîne, sur les consommateurs, dont nous ne serons probablement saisis de l'ampleur que dans les années à venir. Dès lors, que faire ? La mission commune d'information sur les pesticides et leur impact sur la santé, présidée par Mme Sophie Primas et rapportée par Mme Nicole Bonnefoy, a fait de très nombreuses propositions. Les auteurs du texte les ont traduites par la création d'un fonds d'indemnisation dédié, financé par une fraction de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques. Je remercie les auteurs de s'être saisis de cette question face à la carence des gouvernements successifs qui, bien que conscients des enjeux, n'en ont jamais pris la pleine mesure. Je remercie également le rapporteur pour son travail.

notamment, à la nécessité de réformer le système de réparation des victimes de maladies professionnelles en facilitant les démarches de reconnaissance des maladies et en prenant en compte plus efficacement les avancées scientifiques. Il était également question de gestion et d'uniformité des procédures. J'y reviendrai. Aujourd'hui, et nous en sommes tous d'accord, le système d'indemnisation n'est pas à la hauteur et trop de gens sont dans le désarroi. Les constats effectués par la mission en 2012 sont malheureusement toujours d'actualité : les tableaux de maladies sont trop peu nombreux, les critères d'accès à l'indemnisation, trop rigides, les informations concernant les pathologies et leur lien avec l'exposition aux pesticides, insuffisantes. Le financement repose uniquement sur la solidarité nationale, sans pour autant garantir une équité de traitement entre les personnes concernées. Il faut donc le faire évoluer. Je ne pense pas qu'il soit pour autant opportun de créer un fonds. Je ne pense pas non plus que le financement prévu aujourd'hui soit suffisant : c'est d'ailleurs l'avis même du rapporteur, qui indique que cette taxe sera amenée à évoluer. Je crois enfin que la caisse centrale de la MSA ne souhaite pas assumer la gestion d'un tel fonds. Ces constats conduiront la majorité de notre groupe à s'abstenir sur ce texte. Cependant, nous ne nous opposerons pas à cette proposition de loi, car elle a le mérite d'obliger le Gouvernement à agir, et à agir vite. Créer un fonds dédié irait à l'encontre de la ligne de conduite que nous souhaitons voir respectée sur la simplification et la rationalisation de notre système de protection sociale. Les mécanismes existent, il faut les faire évoluer, pas en ajouter de nouveaux. L'indemnisation des victimes de pesticides est possible en cas de reconnaissance d'une maladie professionnelle et se fonde sur des tableaux qui recensent ces pathologies. Ces tableaux doivent pouvoir être complétés plus rapidement sur la base d'informations fiables et permettre une indemnisation plus étendue. Nous pensons d'abord aux agriculteurs. Mais les jardiniers, cantonniers, employés d'entreprises de produits phytopharmaceutiques sont également concernés et ne doivent pas être oubliés. Les critères d'indemnisation doivent, en effet, prendre en compte cette diversité d'usages et d'usagers. Il faut également prévoir un financement pérenne et une gouvernance efficace. Le financement repose aujourd'hui uniquement sur la solidarité nationale. La proposition de loi prévoit un financement par la taxe sur les produits phytopharmaceutiques. N'est-il pas plus juste de prévoir un financement mixte ? L'industrie doit participer, mais cela ne saurait être suffisant pour garantir une indemnisation complète.

nous ont tous bouleversés au plus haut point. Malheureusement, force est de constater que cette proposition de loi n'y répond que partiellement, les enjeux étant beaucoup plus importants. C'est au Gouvernement d'agir avec tous les moyens dont il dispose et avec le soutien du Parlement, qui travaille sur ce sujet depuis de nombreuses années. Il me semble dès lors plus efficace d'aborder cette question dans le cadre du prochain PLFSS, dans quelques mois. lors de la discussion du PLFSS pour 2018, ce qui était naturel, car vous veniez de prendre vos fonctions. Il faut maintenant vous engager résolument à faire évoluer l'indemnisation des victimes de ces produits pour la rendre plus efficace, plus juste et pérenne. La question de l'indemnisation n'est qu'une facette d'une problématique beaucoup plus générale. Il est en effet temps de revoir notre système de production, car notre agriculture et, surtout, nos agriculteurs sont à bout de souffle. Comment expliquer que ceux qui nourrissent les autres ne puissent même plus vivre de leur activité ? Nos différents modes de production doivent tendre chaque jour davantage vers un modèle plus durable. Il n'est plus possible aujourd'hui d'avoir recours à des produits dont les conséquences sur la santé et l'environnement sont si néfastes. Prévoir des protections pour les usagers ne sera jamais suffisant. Il faut développer de nouveaux produits plus naturels, plus sûrs. Nous plus naturels, plus sûrs. Nous ne pourrons pas éternellement réparer. Il faut être capable de changer le système, d'anticiper. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues 1 000, c'est le nombre de substances actives présentes sur le marché. La France est championne européenne des achats de produits phytosanitaires avec, sur les cinq dernières années, une moyenne de 66 000 tonnes par an. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que ces produits ont une influence néfaste sur la santé, et d'abord sur celle des utilisateurs, dont je suis. En effet, être paysan aujourd'hui, c'est s'exposer à une multitude de produits dangereux. Et s'il est facile de nous accuser d'être les premiers pollueurs, il faut savoir que nous sommes, d'abord, les premières victimes. Entre 2013 et 2016, 236 maladies, soit 59 en moyenne par an, ont été reconnues et ont reçu un premier paiement au régime agricole. Pour comprendre pourquoi nous les utilisons quand même, il faut comprendre le travail de la terre. Car nous ne sommes pas des fous inconscients ! Les agriculteurs ont toujours fait appel à des substances pour éradiquer les nuisibles : insectes, champignons, etc. Comment en sommes-nous arrivés à une surenchère de consommation de produits La crise agricole qui nous a frappés de plein fouet et qui continue de faire des ravages sur fond de guerre des prix les plus bas, de différences de droits sociaux, de différences de contexte juridique, notamment pour les produits phytosanitaires, a incité les agriculteurs à favoriser les produits de synthèse nettement moins chers et plus faciles d'utilisation, quelles que soient les conditions atmosphériques. Pour tirer un revenu annuel moyen de 13 500 euros, l'agriculteur essaye de réduire ses coûts de production. C'est logique. À cela s'ajoute un autre point négatif, connu des seuls utilisateurs. L'agriculteur doit se protéger avec une combinaison, des gants, des bottes et un masque, mais il ne les met pas toujours. quand vous êtes dans la cabine d'un tracteur où il fait 40 degrés, vous pouvez imaginer la situation ... Bref, il faut revoir totalement le problème à la base. Les pouvoirs publics doivent obliger les fabricants à innover, à inventer des produits efficaces sans risque pour les utilisateurs et les populations. En attendant, il faut adapter le dosage des produits actuels au stade végétatif de la plante, ce qui engendrera une diminution notable de la consommation des produits Investir dans la recherche, c'est à terme économiser les deniers publics, puisque nous sommes aujourd'hui réunis pour traiter de l'indemnisation des victimes de ces produits, qui, je le rappelle, sont vendus en toute légalité alors que leurs incidences sont notoires dans l'alimentation, l'eau de consommation, l'air et les sols. Cette proposition de loi d'indemnisation des victimes de produits phytosanitaires est un vrai pas en avant, et je remercie son auteur, Nicole Bonnefoy. Il faut, enfin, continuer à repenser notre modèle agricole. Le plan de route d'une agriculture durable établi en 2014 la loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt fixe le cap d'une réduction de produits phytosanitaires. Je suis viticulteur. La viticulture, qui représente 8 % de l'agriculture française, utilise 20 % des produits phytosanitaires. Pourtant, certains se sont lancés avec audace dans l'agriculture bio ou raisonnée, privilégiant la biodiversité. Il faut continuer à les encourager pour que, demain, leur réussite fasse des émules. C'est pourquoi je m'investis dans le dossier des cépages résistants, aux côtés de la filière et de l'INRA. Ces cépages, qui résistent sans traitement à l'oïdium et au mildiou, les deux maladies les plus répandues dans la culture de la vigne, sont l'avenir de notre viticulture, car ils répondent à la fois aux enjeux économiques et sanitaires. Accuser, jeter l'opprobre ne fait pas avancer. Il faut inciter les agriculteurs à d'autres modes de production, et toujours expliquer les enjeux. Ceux de santé publique doivent être notre unique leitmotiv. Nous ne pouvons être responsables de maux que nous sommes les premiers à subir. Pour les victimes, à l'échelle d'une vie, le temps judiciaire, c'est du temps perdu.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes bien peu nombreux pour discuter d'une affaire importante, permettez-moi néanmoins de féliciter chaleureusement nos collègues Nicole Bonnefoy,

à l'ordre du jour de nos discussions. Ce texte puissant, équilibré et éminemment d'actualité me semble aller au-delà de la simple indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques. Ouvrir un droit à l'indemnisation, c'est reconnaître une faute, notamment celle d'avoir autorisé l'utilisation de produits dangereux, voire mortels,

à savoir la contamination volontaire au chlordécone. Pendant plusieurs décennies, l'État et l'Europe, à travers leurs agences et leurs services, ont

qui a autorisé l'utilisation de ce pesticide jusqu'en 1990, alors même que sa toxicité était connue depuis les années soixante-dix, grâce notamment aux rapports Snegaroff de 1977 et Kermarrec de 1980. Outre ce blanc-seing octroyé aux industriels et producteurs pour poursuivre leur funeste entreprise, l'État a sciemment commis la faute inexcusable d'accorder une dérogation exceptionnelle de trois ans supplémentaires à nos industriels et commerçants pour l'utilisation de ce pesticide, déjà interdit depuis 1976 aux États-Unis. Deuxièmement, l'État, sous couvert de l'Europe, a appuyé la demande des industriels pour relever à deux reprises, en 2008 et 2013, les limites maximales de résidus, seuil au-delà duquel la commercialisation des denrées alimentaires est interdite.

par son attentisme, l'État n'a pas pris les décisions à même de répondre à la psychose collective qui s'est emparée de nos compatriotes. Les études épidémiologiques, au nombre de quatre me semble-t-il, non actualisées et non répétées, sont insuffisantes et parcellaires. Les plans chlordécone I, II et III évoqués par la ministre sont sous-dotés et sous-consommés. La traçabilité des produits est inopérante, les actions de prévention demeurent confidentielles

totalement intégrée, et c'est la raison pour laquelle un plan sur les phytosanitaires est en cours de discussion. La feuille de route est d'ores et déjà rédigée. Elle vise évidemment à réduire l'exposition à la fois des travailleurs exposés et des populations vulnérables. Elle tend aussi à l'éviction,

la reconnaissance des maladies faite au cas par cas par les comités régionaux de reconnaissance. Ces comités sont trop hétérogènes et ne tiennent pas forcément compte des données de la science. Un travail sera fait pour leur proposer des référentiels de prise en charge et une harmonisation des pratiques pour qu'il n'y ait plus d'aléa ou d'arbitraire.

Je serais ravie de pouvoir rendre compte de l'évolution de ce plan devant vous et devant la commission des affaires sociales. La discussion

certaines vérités qui me semblent très largement partagées par les Martiniquais et les Guadeloupéens. Prétendre que les organochlorés ne peuvent pas figurer dans le périmètre de définition des produits phytopharmaceutiques au motif

soit remis au goût du jour à travers cette proposition de loi extrêmement intéressante. Madame la ministre, je fais partie de ceux qui ont été très déçus par vos propos.

personnes exposées. La parole est à Mme Catherine Conconne, sur l'article. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, c'est avec grand plaisir que je participe aujourd'hui à ce débat sur la proposition de loi de ma collègue Nicole Bonnefoy et du groupe socialiste. Ce texte ne saurait mieux tomber. En effet, depuis le 26 décembre dernier, la presse antillaise s'est fait l'écho de préoccupations relatives à une augmentation des limites maximales de résidus de chlordécone aux Antilles, les fameuses LMR, à la suite de l'étude « Kannari de l'ANSES sur l'exposition de nos populations les denrées alimentaires. Je vous rappelle notre triste histoire avec le chlordécone, dont mon collègue Victorin Lurel vient de parler

Ce texte vise tout d'abord à protéger et défendre les malades des pesticides, au premier rang desquels les agriculteurs. Je me réjouis des travaux du Sénat, qui s'attellent aujourd'hui à améliorer la réparation du préjudice que subiront plusieurs générations. Accepter d'indemniser

Cet argument n'est absolument pas recevable, madame la ministre. On ne peut pas dire aux victimes de se débrouiller dans des actions en réparation devant les tribunaux civils, car, vous le savez bien, la puissance des avocats des industriels est telle

ce lien de causalité et, en conséquence, demandera la réparation intégrale. C'est cela, la justice, madame la ministre

D'abord, les risques sur la santé des expositions environnementales ne sont malheureusement pas bien connus et sont insuffisamment documentés sur le plan scientifique. Ensuite, un tel dispositif d'indemnisation serait déresponsabilisant, en particulier à l'égard des industriels. Même si je suis d'accord avec vous, les effets sur la santé des produits phytopharmaceutiques en général font l'objet d'un consensus scientifique concernant des expositions professionnelles. Il me semble plus pertinent de renforcer l'indemnisation dans le cadre du système préexistant des accidents du travail et des maladies professionnelles, et de donner la priorité absolue à la prévention des risques liés à ces produits. C'est dans cette optique que le Gouvernement compte renforcer l'effort de recherche, ... Avec quels moyens ? ... afin de mieux connaître les liens entre pathologie et exposition,

Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'agriculture ne peut valablement établir une liste des pathologies mentionnées aux 2° et 3° du présent article sans un avis préalable d'experts médicaux compétents-

Je profite de cette prise de parole pour continuer à répondre aux arguments de Mme la ministre.

de la proposition de loi prévoit une subrogation dans les droits. Rien n'empêche au demandeur, au patient, de demander réparation au responsable, employeur, industriel.

Joël Labbé, sur l'article. S'il semble logique de confier de manière formelle la gestion du fonds d'indemnisation à la MSA, il faudra être très vigilant sur la composition du conseil de gestion, afin que celui-ci soit

pollueurs, « indemnisateurs »- cela fait un peu beaucoup -, c'est-à-dire juge et partie, cherchant à tout prix- on sait qu'ils fonctionnent ainsi -à empêcher la reconnaissance des pathologies dans l'espoir d'amoindrir leur contribution financière à ce fonds. à ce fonds. La parole est à Mme Catherine Conconne, sur l'article. Je tiens également à saluer l'amélioration de l'expertise pour la détermination des liens entre exposition et pathologie. La création de ce fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques, assorti d'une commission médicale autonome, me semble très efficace. Aujourd'hui, l'évaluation des risques est permanente, et c'est avec exactitude que l'on suit l'évolution entre exposition et effets potentiels sur la santé humaine. Cette commission aura pour

sans protection. Pour ma part, j'ai eu la chance d'être extrêmement sensible à ces produits et de m'être protégé très tôt. Mais on ne peut pas se protéger totalement. J'ai régulièrement été affecté par des vomissements,

Merci, monsieur le rapporteur ! Quel est l'avis du Gouvernement ?

à identifier des effets à moyen et à long terme, car les effets à court terme du chlordécone sont connus. Ayant aussi été vice-présidente du Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC,

méthodologique, c'est excessivement compliqué, car il s'agit d'expositions très anciennes qui touchent l'ensemble de la population. Aussi, c'est un problème scientifique qui persiste aujourd'hui, monsieur Lurel. Sachez à quel point j'ai été mobilisée et je continue l'être en ma qualité de ministre pour essayer de mieux comprendre les effets à moyen et long termes du chlordécone sur vos populations.

Cette liste est, me semble-t-il, beaucoup plus longue que celle des produits pour lesquels, après vérification, aucune relation de cause à effet

médical, voire, comme le prévoit un amendement de nos collègues du groupe Les Républicains, le secret industriel et commercial. Ce dernier peut en effet empêcher des victimes de prouver leur intoxication,

de caractériser le lien entre les expositions et les pathologies, de garantir le secret médical ainsi que le secret industriel et commercial. Comme dans le cas du conseil de gestion du fonds, la composition de la commission médicale sera essentielle pour garantir son impartialité, sa transparence et sa compétence médicale. En effet, nous savons aujourd'hui les dégâts que peuvent engendrer les conflits d'intérêts dans les questions de santé publique. La parole

C'est pourquoi je me réjouis que cette proposition de loi facilite le parcours de reconnaissance de la maladie professionnelle. Ce texte vise à mettre un terme à cette autre injustice faite aux victimes que constituent la longueur et la difficulté des procédures visant à faire reconnaître le lien entre exposition et pathologie et à obtenir une indemnisation. Cette procédure simplifiée, uniformisée et plus juste pour les malades permettra un traitement efficace et impartial des préjudices subis par nos professionnels exposés. L'introduction en commission des affaires sociales de la présomption de causalité, en remplacement de la justification du lien direct, permettra un accès facilité aux soins. Elle favorisera également un changement de mentalité pour et autour des victimes, pour lesquelles la justification de l'existence d'un lien de cause à effet entre exposition et pathologie, qu'elle était contraignante à évaluer, tenait du chemin de croix, si ce n'est du parcours du combattant

La commission médicale doit disposer de la possibilité de procéder, ou de faire procéder, à toute expertise et investigation utiles à l'examen du lien direct entre l'exposition aux produits phytopharmaceutiques et la pathologie alléguée. De plus, les données échangées au sein de cette commission doivent

nous demandons la création d'une commission scientifique indépendante, dont les membres ne seraient pas rémunérés. J'ose le dire devant cette auguste assemblée, puisque le gage est presque levé : c'est l'astuce que nous avons trouvée pour contourner l'article 40

son incidence sur la pollution des sols et des rivières en Guadeloupe et en Martinique. Je le répète : il est très clair que le chlordécone et le paraquat sont des produits phytopharmaceutiques. qu'ils ne soient plus utilisés n'oppose aucun obstacle à la réparation des dommages subis. Il va de soi que l'utilisation de ces produits et ses conséquences sur la santé sont incluses

que c'est le tabac qui a déclenché le cancer du poumon. Cela étant, le lien de causalité est très probable. En conséquence- c'est la jurisprudence en la matière -, la certitude juridique n'exige pas la certitude scientifique.

fonds. Quel est l'avis de la commission ?

Le présent amendement a pour objet d'inciter les utilisateurs de tels produits à respecter les conditions d'utilisation figurant sur les étiquettes et, ainsi, d'éviter l'aggravation de leur état de santé.

253-8-2 du code rural et de la pêche maritime, versée annuellement, ne paraît pas nécessaire lorsque le fonds est suffisamment alimenté pour indemniser les victimes. Aussi, le présent amendement vise la modulation de la fraction de la taxe perçue par le fonds par le fonds en fonction de ses besoins financiers et des sommes perçues au titre des recours subrogatoires en application de l'article 6 de cette proposition de loi. Quel est l'avis de la commission ? La taxe actuellement collectée sur les produits phytopharmaceutiques finance les actions de phytopharmacovigilance déployées par l'ANSES.

concerne la totalité des denrées alimentaires, qu'elles relèvent des circuits contrôlés ou non contrôlés. Tel est le travail que nous aurons à faire ensemble dans les mois qui viennent. Merci, madame la ministre ! Je mets aux voix l'article 8. L'amendement

Monsieur le président, madame la ministre,

Mais je crois en vous. Je crois en votre sincérité. Je dirai même que l'on vous sent touchée par ce sujet.

bousculer ainsi l'inertie des pouvoirs publics. Pour ma part, je suis également heureux d'avoir pris part à ce débat en commission et dans l'hémicycle, l'hémicycle, avec mes collègues de la Guadeloupe et de la Martinique, pour plaider la cause de nos populations, s'agissant de la question du chlordécone et du paraquat. Comment pouvait-il en être autrement ?

Je sais quel sera votre sentiment final en la matière, mais je vous incite vraiment à entendre la voix de la Haute Assemblée afin de défendre celles et ceux qui croient en nous

demande, madame la ministre, de faire en sorte qu'il en soit ainsi, afin de faire avancer la reconnaissance des maladies et leur réparation intégrale.

mais aussi ceux qui nous ont demandé de les représenter dans la Haute Assemblée ne comprendraient pas que nous ne votions pas ce texte à deux mains, à dix mains, à mille mains

ces oeufs du pays sont impropres à la consommation. Pour ces populations, nous sommes très fiers, nous, Guadeloupéens et Martiniquais en particulier, citoyens les plus touchés de la République par les produits pesticides, de voter

oui. Il ne faut intervenir ni trop tard- nous en savons les conséquences -ni trop tôt. Or il n'est pas trop tôt, car la connaissance scientifique, même si elle est encore en mouvement, est déjà bien établie. Le Sénat

Dans la discussion générale, la parole est à M. Jean-Yves Leconte, auteur de la proposition de loi. Monsieur

pour établir une solidarité entre les Français vivant hors de France en termes d'assurance maladie. On y adhère volontairement, elle fonctionne dans le cadre des règles de la sécurité sociale et elle assure les remboursements de prestations réalisées dans le monde

l'étranger. Le dispositif construit dans les années 1980 n'est plus adapté aux personnes qui ont des contrats locaux, à celles qui se rendent à l'étranger pour créer une entreprise ou qui s'installent pour y vivre sans être détachées par une grande entreprise. Les adhérents individuels sont aujourd'hui en effet

La CFE n'étant pas un régime obligatoire, elle rencontre des difficultés à évoluer au regard de ces exigences de l'expatriation et du monde. Et puis il y a l'Europe. Les textes des années 1980 ont été jugés contraires au principe d'égalité de traitement des ressortissants de l'Union européenne. Par conséquent, depuis

des prestations d'assurance maladie à l'ensemble des ressortissants européens qui souhaitent s'affilier à la Caisse des Français de l'étranger. Aujourd'hui, l'état des lieux est le suivant : l'offre tarifaire est très complexe,

aujourd'hui. Compte tenu de ces éléments qui bloquent le développement de la Caisse des Français de l'étranger, nous constatons une augmentation inquiétante de l'âge moyen de ses assurés qui pourrait un jour remettre en cause son équilibre. Il est donc urgent

s'inspire d'amendements qui ont été déposés l'année dernière par Christophe-André Frassa et moi-même lors de la discussion d'autres projets de loi, ainsi que d'une proposition de loi de Joëlle Garriaud-Maylam. Je salue également le travail du rapporteur, Yves Daudigny,

L'idée générale de cette réforme est d'unifier les modes de calcul des cotisations d'assurance maladie-maternité et invalidité pour que l'ensemble des adhérents, anciennement catégorisés en salariés, travailleurs indépendants, pensionnés ou étudiants, cotisent en fonction non plus de ces catégories

et à la situation globale du marché de la santé dans le monde. Depuis deux ans, la Caisse a fait le maximum pour se moderniser et pour répondre au mieux aux besoins, mais elle ne peut pas aller plus loin sans modification législative. Cette proposition de loi répond à cette exigence.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, pour l'observateur familier de la sécurité sociale, la Caisse des Français de l'étranger, ou CFE, est un objet de curiosité et d'intérêt. Conçue comme le prolongement de la sécurité sociale à l'étranger pour les expatriés, elle en reprend certaines caractéristiques, mais elle s'inscrit dans un tout autre environnement, en concurrence avec d'autres acteurs. acteurs. Jean-Yves Leconte a exposé les motifs qui ont conduit nos collègues représentant les Français établis hors de France à travailler, avec la Caisse, à une réforme de son cadre législatif que le Sénat examine cet après-midi. Je n'y reviendrai pas. J'indiquerai en revanche quels ont été l'état d'esprit de la commission des affaires sociales et ses principales observations. Afin de bien identifier les enjeux de ce texte et ses conséquences concrètes pour nos compatriotes établis à l'étranger, j'ai souhaité rencontrer les représentants des deux principales associations des Français de l'étranger. Je remercie Claudine Lepage,

une grande convergence de vues sur la nécessité de revoir l'offre tarifaire de la Caisse et d'améliorer la lisibilité de ses prestations. Saisie de ce texte, la commission des affaires sociales a confirmé ces objectifs. Leur atteinte suppose qu'une plus grande capacité d'initiative soit donnée au conseil d'administration de la Caisse. Ces modifications législatives sont relativement urgentes puisque, sur le fondement de décisions du conseil d'administration intervenues en juin 2016, la Caisse a commencé à proposer de nouveaux produits une offre pour les soins en France et, très récemment, une offre en direction des jeunes. Elle mène également, sur le volet de ses prestations, une expérimentation en Thaïlande qui pourrait être généralisée. La commission des affaires sociales a souhaité préserver les équilibres issus des travaux menés par nos collègues avec la Caisse. La réécriture du texte à laquelle elle a procédé ne doit pas occulter cette volonté. La commission a tiré les conséquences, dans la structure du chapitre concerné du code de la sécurité sociale, du changement d'approche induit par la proposition de loi, d'une logique de catégories d'adhérents- salariés, travailleurs indépendants, pensionnés, étudiants, chômeurs ... -à une logique de risques couverts- maladie-maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles.

limité les modifications apportées au droit en vigueur à l'adaptation de la composition du conseil d'administration, à la suppression des différentes catégories d'adhérents, à l'actualisation des conditions d'éligibilité et à l'obligation de la parité dans la constitution des listes. Il lui semble que ces modifications, sans répondre à l'ambition initiale du texte, peuvent réunir un consensus. Le conseil d'administration a été renouvelé récemment

Le Sénat aura sans doute à examiner de nouveau la question de la gouvernance de la CFE. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, telles sont les principales observations qu'appelle la proposition de loi à réforme de la Caisse des Français de l'étranger que la commission des affaires sociales vous demande d'adopter dans la rédaction issue de ses travaux. La parole

En effet, si depuis près de quarante ans la CFE s'est imposée comme une référence, elle agit aujourd'hui dans un cadre contraint, et donc sans les outils pour répondre aux attentes d'une communauté française à l'étranger qui ne cesse de s'agrandir. D'abord, les attentes des Français de l'étranger en matière de couverture sociale sont importantes. Ainsi, selon un très récent baromètre sur la protection sociale des expatriés, 75 % des Français de l'étranger interrogés jugent important de garder le lien avec le système français de protection sociale, et près de la moitié- 49 % -, déclarent que la protection sociale « à la française » fait partie de ce qui leur manque le plus à l'étranger. Cette demande provient d'une communauté française à l'étranger qui continue de s'accroître dans des proportions très importantes. Aujourd'hui, près de 1,8 million de Français sont inscrits au registre des Français établis hors de France, et l'on estime entre 2 et 2,5 millions le nombre total de Français établis hors de notre territoire de manière permanente ou quasi permanente. Pour accompagner la mobilité des Françaises et des Français et leur garantir une continuité de la protection sociale, nous disposons actuellement de deux outils. D'abord, mais je ne m'étendrai pas sur cette possibilité, cette continuité est garantie les conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par la France et les règlements européens de coordination. La coordination des législations de sécurité sociale permet ainsi d'assurer que les droits acquis dans deux ou plusieurs systèmes soient reconnus et valorisés dans chacun des systèmes de protection sociale. Le second outil, qui nous occupe aujourd'hui, est la CFE et les garanties qu'elle propose. Il peut intervenir en complément de la coordination en cas de couverture locale insuffisante, ou s'imposer comme l'unique choix pour l'expatrié à défaut d'accord conclu avec la France. Or les réponses fournies actuellement par la Caisse ont été conçues il y a très longtemps, dans un autre contexte, et ne sont plus du tout adaptées. L'offre, en particulier en matière de santé, s'est compliquée et est devenue peu lisible. Les garanties sont souvent perçues comme offrant une couverture trop limitée Près de quarante ans après sa création, la Caisse doit donc se moderniser pour éviter un trop grand décalage avec le nouveau visage de l'expatriation et pour mieux répondre aux attentes des Français de l'étranger. C'est dans cette perspective que le Gouvernement apporte son soutien à cette proposition de loi, notamment au texte de la commission. Les évolutions aujourd'hui proposées doivent permettre d'améliorer la protection sociale de nos expatriés selon plusieurs axes : une meilleure lisibilité des garanties à travers une offre plus claire, une grille tarifaire rénovée pour la couverture maladie et une prise en charge des soins de santé à l'étranger plus adaptée. La proposition de loi prévoit également de permettre à la Caisse des Français de l'étranger de sortir du statut dans lequel elle est enfermée, afin qu'elle puisse nouer des partenariats avec des courtiers et des assureurs tout en restant connectée à la protection sociale française. Je n'oublie pas le volet gouvernance, dont les ajustements aujourd'hui envisagés contribueront à la bonne représentation au sein du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger, ne serait-ce qu'en termes d'exigence de parité. Cette évolution s'inscrit d'ailleurs dans le mouvement de modernisation engagé par les caisses de sécurité sociale. Globalement, ces évolutions devront permettre de mieux répondre aux attentes de nos concitoyens et recueillent en conséquence le total soutien du Gouvernement.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous abordons l'examen de la proposition de loi de nos collègues socialistes dans le contexte d'une éventuelle réforme de la représentation des Français de l'étranger, avec la tenue de consultations et l'ouverture probable d'un chantier sur ce sujet. Aussi ce texte intervient-il peut-être un peu trop tôt.

Pourtant, il faudra bien un jour tirer les conséquences de la loi de 2013 qui a réduit le nombre de membres de l'AFE, l'Assemblée des à 90 et instauré leur élection par les conseillers consulaires dans le but d'une meilleure proximité des expatriés avec leurs élus. Ces dispositions induisent une réduction mécanique du corps électoral pour l'élection des représentants de la Caisse. C'est pourquoi il faut bien reconnaître l'intérêt de l'élection du conseil d'administration par les 500 conseillers consulaires. Outre l'élargissement du corps électoral, une telle modification permettrait également la suppression d'un degré d'élection. Mais visiblement, le rapprochement des assurés de leurs représentants n'est pas encore à l'ordre du jour. Je ne m'étendrai pas plus Je rappellerai tout de même que, en 2015, la proposition de loi de notre collègue Jean-Yves Leconte sur ce thème avait été rejetée, certains arguant qu'il fallait attendre les conclusions de l'enquête de l'Inspection nous y voilà ! Le rapport a été rendu quelque temps après, la même année. Plus rien ne s'oppose à cette réforme, à moins que des enjeux de pouvoirs ne génèrent toutes ces tergiversations et lenteurs La principale innovation du texte tel qu'il résulte des travaux de la commission réside donc dans son premier volet relatif à la réforme de l'offre tarifaire pour l'assurance maladie. Cette réforme était annoncée depuis 2015, date à laquelle l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales ont mené une réflexion globale sur l'évolution des missions et de la gestion de la Caisse des Français de l'étranger. Leur rapport mettait alors en exergue la nécessité de rénover la politique commerciale et l'offre tarifaire de la Caisse, afin de les adapter aux nouvelles formes et aux nouveaux parcours de l'expatriation. Selon les auteurs de la proposition de loi, la Caisse proposerait en effet plus de 600 tarifs modulés en fonction de l'âge des assurés, du niveau de revenus, du paiement ou non des cotisations par une entreprise, ou encore de la catégorie d'adhérents. Dans un contexte concurrentiel où la plupart des organismes d'assurance maladie ont développé une offre de couverture à l'expatriation, il est essentiel d'améliorer la lisibilité des prestations de la Caisse et de renforcer son action auprès des jeunes actifs. Le rapport de l'IGAS et de l'IGF relevait également une incompatibilité avec les règles européennes. L'adhésion à la Caisse ne saurait en effet être réservée aux seuls Français. Il aura donc fallu attendre plus de deux ans pour entreprendre la réforme préconisée en juillet 2015. Aussi, je salue l'initiative de nos collègues représentant les Français établis hors de France du groupe socialiste qui ont travaillé avec la Caisse à une évolution de la base législative régissant son offre. Créée en 1984 dans le prolongement de la Caisse des expatriés, la CFE est devenue au fil des années un acteur majeur de la protection sociale des Français de l'étranger et couvre plus de 200 000 personnes à travers le monde. Il était donc urgent d'entamer cette réforme, d'adapter la Caisse à son temps, de la tourner vers l'avenir » pour reprendre les termes de notre collègue Jean-Yves Leconte. Le nombre considérable de Français travaillant aujourd'hui à l'étranger nous semble justifier que notre assemblée s'en préoccupe. Je tiens à saluer l'excellent travail du rapporteur, qui a réécrit le dispositif tout en préservant son esprit. Il permettra de passer d'une logique de catégories d'adhérents à une logique de risques couverts. C'est une bonne chose.

Le conseil d'administration a été renouvelé en 2015 et c'est maintenant M. Alain-Pierre Mignon qui préside à sa destinée avec dynamisme. Ses projets pour la CFE sont à l'origine de la proposition de loi dont nous discutons. La CFE transpose très largement les règles de gestion de la sécurité sociale française moyennant quelques adaptations. Ainsi, les règles d'adhésion à la CFE reproduisent fidèlement les différents statuts que connaît la sécurité sociale française- salarié, non-salarié, étudiant, retraité, inactif -avec leurs spécificités. Il en est de même pour les règles de prise en charge des soins, avec la complexité que représente la transposition à l'étranger de ces règles de gestion. Pendant de nombreuses années, la CFE s'est développée en accompagnant le développement international des entreprises dans le contexte de la mondialisation. Elle a également pris en charge une part croissante de Français s'expatriant à titre individuel- jeunes à la recherche d'un premier emploi, retraités, entrepreneurs tentant une nouvelle aventure en milieu de carrière La Caisse a atteint son apogée en termes de risques couverts en 2014. Au début de l'année 2016, la CFE a connu une évolution significative après le renouvellement de son conseil d'administration. Le bureau du conseil a mené un audit approfondi de la Caisse et a constaté une diminution du nombre d'assurés, amorcée depuis 2014, couplée à un certain défaut d'attractivité vis-à-vis des jeunes. Ce diagnostic qui aurait pu, à terme, menacer l'équilibre de la Caisse, l'a conduite à envisager des mesures nouvelles, qui justifient les évolutions législatives sur lesquelles nous allons nous prononcer. La Caisse a souhaité lancer une réforme des cotisations selon une logique tarifaire assise sur l'âge et la composition de la famille de l'assuré. Elle propose d'offrir deux types de produits. En premier lieu, le produit FrancExpat Santé, qui prend en charge uniquement les soins en France, a été lancé au début année. Fort du constat que 50 % des remboursements sont liés à des soins en France, ce produit s'adresse essentiellement aux Français résidant dans des pays dans lesquels il existe un système de protection sociale obligatoire rendant l'adhésion à la couverture mondiale de la CFE moins utile. En deuxième lieu, la proposition de loi prévoit une réforme globale, rendant plus simple et plus lisible le dispositif tarifaire qui serait arrêté par le conseil d'administration de la CFE en fonction de l'âge et de la composition de la famille de l'assuré. permettra ainsi à la Caisse de prendre en charge les soins dans le monde entier en se substituant au dispositif actuel. Le produit JeunExpat Santé, lancé en juin 2017, constitue une première étape réussie de cette ambitieuse réforme. Cette réforme structurelle ne remet pas en cause les fondements de caisse de sécurité sociale de la CFE et les valeurs de solidarité liées à son objet social. Il existe déjà un dispositif de « catégorie aidée » qui permet la prise en charge d'une partie des cotisations pour les Français disposant de ressources inférieures à un certain seuil par le budget d'action sociale de la Caisse. Ce dispositif serait renforcé dans le cadre de cette réforme. La Caisse souhaite également mieux définir les garanties qu'elle offre à ses clients et assurer un plus large accès en tiers payant dans un nombre beaucoup plus important d'établissements de soins. Elle a, dans cette optique, lancé une expérimentation en Thaïlande. Il s'agit de la prise en charge en tiers payant des frais hospitaliers à hauteur d'un taux forfaitaire, en lien avec un partenaire disposant d'un réseau de soins. Avec cette réforme, la Caisse pourra désormais adapter les règles de prise en charge des soins pour les rendre plus lisibles et plus simples à gérer et garantir ainsi un meilleur service sans s'écarter significativement des tarifs pratiqués en France pour des soins analogues. En effet, il n'est pas question pour elle de sortir de son rôle de caisse de sécurité sociale de base. En revanche, la loi lui permettra de conclure des partenariats avec des assureurs complémentaires pour offrir à ses clients une prise en charge complète des soins qu'ils engagent. Cette réforme propose de donner à la CFE une certaine latitude pour adapter l'offre tarifaire et les garanties en fonction de l'évolution des besoins de nos compatriotes expatriés. Elle constitue un acte de confiance envers le conseil d'administration de la Caisse. Cette souplesse conférée au conseil d'administration interviendra bien entendu sous le contrôle des pouvoirs publics. En effet, les décisions prises par ce conseil dans ce nouveau cadre législatif devront être entérinées par arrêté ministériel. Je remercie Jean-Yves Leconte d'avoir obtenu de son groupe que la présente proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour. Je me suis pleinement investie avec lui, en lien avec d'autres collègues représentant les Français de l'étranger, plus particulièrement Christophe-André Frassa et Ronan Le Gleut, pour que cette réforme transpartisane soit une réussite pour nos compatriotes expatriés. Mes remerciements vont également au rapporteur de la commission, Yves Daudigny, qui a effectué un travail remarquable pour préciser le texte initial. On peut dire que le texte résultant des travaux de la commission est une véritable oeuvre collective à laquelle tous ont travaillé en lien avec le président, le conseil d'administration et la direction de la Caisse. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, le groupe Les Républicains soutient cette proposition de loi. J'espère que le Gouvernement accompagnera cette réforme nécessaire au renforcement de la protection sociale de nos compatriotes expatriés par un avis favorable sur ce texte. En votant ce dernier, nous ferons oeuvre utile pour nos compatriotes expatriés et pour le renforcement de notre modèle social.

essentiel et précieux pour les Français de l'étranger et pour ceux qui souhaitent s'expatrier. Les évolutions récentes, accentuées par la crise économique, se traduisent par une baisse du nombre de salariés bénéficiant d'un contrat d'expatriation- ces salariés constituent le public historique de la Caisse -, et par une augmentation du nombre de personnes recrutées sous contrat

Depuis 2016, un vent de réforme souffle sur la Caisse. Son conseil d'administration a été considérablement modifié à la suite des élections de l'AFE, et sa direction a également changé.

la première priorité concerne les modalités de fixation des cotisations. Les assurances volontaires de la CFE sont trop chères

le profil des assurés apparaît en décalage avec celui des Français établis hors de France. Cette situation est préoccupante, car elle fait peser un risque sur l'équilibre financier de la CFE, qui est aujourd'hui assuré grâce aux adhésions des salariés et des grandes entreprises. Il est donc nécessaire de doter la CFE de nouveaux outils juridiques lui permettant de rééquilibrer sa pyramide des âges et de préserver son équilibre. C'est pourquoi il est proposé d'unifier la grille tarifaire de la Caisse, et de l'articuler autour de la tranche d'âge et de la composition familiale de l'assuré.

doit nous conduire à ne pas modifier le droit en vigueur tant que la réflexion sur la représentation non parlementaire des Français établis hors de France n'a pas abouti. Pour toutes ces raisons, le groupe La République En Marche soutient cet excellent texte. La

pour des personnes effectuant une partie de leur carrière à l'étranger, le plus souvent dans le cadre de contrats d'expatriation avec une prise en charge de la protection sociale par l'entreprise et un retour programmé en France. Sa mission d'origine est d'assurer aux salariés français expatriés une continuité de leur couverture sociale. Les Les expatriés sont libres d'adhérer à la CFE, qui fonctionne uniquement grâce aux cotisations de ses adhérents. Ce modèle connaît aujourd'hui une crise du fait de la baisse du nombre d'assurés en raison de l'augmentation du nombre de contrats locaux. Après un contrat français d'expatrié de trois ans renouvelé une fois, les employeurs proposent souvent aux salariés de passer en contrat local. Le développement des contrats locaux, avec des salaires plus faibles que ceux qui sont octroyés en France, ne permet pas toujours aux expatriés de s'assurer auprès de la CFE. L'enjeu de la proposition de loi que nous examinons est de simplifier un régime qui s'est largement complexifié depuis sa création, comptant notamment autant de régimes tarifaires qu'il y a de catégories d'assurés- salariés, non-salariés, étudiants, inactifs Il y a actuellement 600 tarifs possibles ! Cette explosion du nombre de régimes tarifaires a entraîné une illisibilité et un affaiblissement général de la CFE, déjà soumise à une forte concurrence des complémentaires privées étrangères.

en fonction de l'appartenance à une catégorie d'âge et de la composition familiale de l'assuré volontaire, et, pour les adhérents à faibles revenus, cette cotisation pourra être modulée en fonction du niveau des ressources de l'assuré. Je ne suis pas certaine que la coexistence de deux systèmes avec, d'un côté, une cotisation forfaitaire selon la composition du foyer et, de l'autre, une cotisation modulée selon les revenus de l'assuré soit de nature à améliorer la lisibilité des tarifs de la CFE. Concernant les prestations remboursées à l'étranger par la Caisse des Français de l'étranger, nous pensons indispensable que les expatriés puissent connaître, avant toute consultation ou toute opération, le niveau de prise en charge des soins par la Caisse. Enfin, s'agissant du volet de la gouvernance, nous notons avec satisfaction l'application de la parité entre les hommes et les femmes pour la constitution des listes. Malgré ces remarques constructives, nous soutenons les objectifs poursuivis avec cette proposition de loi, à savoir revitaliser la Caisse des Français de

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le vice-président de la commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues,

Il indiquait que la Caisse, se trouvant dans un contexte de concurrence avec les assureurs privés, avait développé des modalités d'intervention qui tendaient à l'éloigner des organismes de sécurité sociale et à la rapprocher d'un assureur privé. En 2015, une mission conjointe de l'IGAS et de l'IGF a formulé un certain nombre de recommandations, préconisant notamment d'améliorer l'offre tarifaire de la Caisse. Elle mentionnait également la nécessité de mettre les textes régissant les conditions d'affiliation à la CFE en conformité avec le principe communautaire d'égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et communautaires. Faisant suite à ces différentes recommandations, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'articule autour de deux chapitres. Le premier concerne l'offre commerciale et le second la gouvernance. Le premier volet procède à l'unification du mode de calcul des cotisations des différentes catégories d'adhérents, en fonction de leur catégorie d'âge et de la composition de leur foyer. Cette mesure apportera une clarification bienvenue à l'offre commerciale de la CFE et lui permettra de se maintenir dans la compétition. L'ampleur du second volet, bien qu'important, est moindre dans la mesure où il se contente de tirer les conséquences de la suppression des différentes catégories d'assurés pour adapter la représentation au sein du conseil d'administration de la Caisse, dans l'attente d'une réforme plus importante plus importante de la représentation des Français de l'étranger, comme cela a été souligné. Cette proposition de loi devrait permettre à la CFE de se refonder pour continuer d'accompagner nos compatriotes installés hors de France.

Haute Assemblée répond aujourd'hui à une sollicitation du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger qui appelle à une réforme rapide, dans un souci d'adaptation aux nouvelles formes et aux nouveaux parcours de l'expatriation. Cette réforme est un acte salutaire pour répondre à une double problématique : d'abord, celle de l'illisibilité de l'offre tarifaire actuelle, avec plus de 600 offres disponibles ; ensuite, celle du manque d'adaptation à une population grandissante, celle des jeunes expatriés, souvent partis étudier à l'étranger pour de courts séjours. La proposition de loi de notre collègue Jean-Yves Leconte a le mérite de dépoussiérer un système en totale déshérence. Elle satisfait l'attente des Français de l'étranger,

Ce n'est pas une mince affaire ! Un peu moins de 2 millions de nos compatriotes vivent aujourd'hui à l'étranger, une proportion en hausse constante depuis plusieurs années. Partout dans le monde, ces Français nous demandent d'adapter le droit français à leur situation d'expatriés. Il nous faut les entendre, adapter la loi à la spécificité de leur situation, et notre chambre a toujours été à leur écoute. Cette réforme de la CFE prévoit surtout une simplification drastique de l'offre tarifaire de l'assurance maladie volontaire. À l'heure d'une remise à plat de notre système de sécurité sociale, c'est une mesure courageuse et nécessaire pour apporter de la clarté et de la lisibilité à nos compatriotes. À l'avenir, la cotisation volontaire sera déterminée en fonction des tranches d'âge et de la composition familiale, quel que soit le statut de l'adhérent et quelle que soit la nationalité des membres de sa famille. Cette petite révolution mérite d'être saluée. Dans un même élan de simplification, la proposition de loi prévoit une prise en charge en fonction du pays où les soins sont prodigués, avec une couverture en pourcentage du coût des soins. Cette adaptation à la diversité des pays est salutaire pour notre modèle de sécurité sociale. Elle apporte davantage de liberté à notre système de couverture médicale et ne retient plus captive la CFE de normes françaises totalement déconnectées des tarifs pratiqués à l'étranger. Dans un souci de respect de la législation européenne, la proposition de loi supprime enfin la condition de nationalité pour adhérer à la CFE. Dans la pratique, cette évolution de notre droit répond à une situation de fait, déjà tolérée par la CFE, puisque la Caisse accepte les adhésions des ressortissants des États membres de l'Union européenne et de pays tiers aux assurances volontaires. Cette mesure devrait donc rapidement se mettre en place. Permettez-moi, avant de conclure, de dire quelques mots sur la réforme de la gouvernance de la CFE. Celle-ci me semble essentielle pour prendre en compte la réforme de juillet 2013 relative à la représentation des Français de l'étranger. Je déplore simplement que nos collègues de la commission aient supprimé la référence au vote par correspondance électronique lors de l'examen de cette proposition de loi. Dans notre effort de simplification du droit, nous ne devons pas manquer de relever le défi

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, j'ai bien compris le message : je serai brève. Je me réjouis que le Sénat examine de nouveau une proposition de loi relative à la protection sociale des Français établis hors de France, sujet éminemment important pour nos compatriotes résidant à l'étranger. Il y a un peu plus de deux ans, nous étions déjà réunis dans cet hémicycle pour débattre d'une proposition de loi visant à réformer la gouvernance de la Caisse des Français de l'étranger, mais, malheureusement, la majorité sénatoriale avait fait le choix de s'opposer Aujourd'hui, la présente proposition de loi comporte deux volets complémentaires et indispensables pour faire entrer pleinement la CFE dans le XXI siècle et l'adapter- enfin ! -à l'évolution de la représentation politique des Français établis hors de France et à la réalité de l'expatriation. Il nous a en effet paru indispensable d'ajouter un volet commercial au texte initial. Créée il y a quarante ans, la Caisse des Français de l'étranger doit nécessairement s'adapter aux changements que connaît l'expatriation et à l'évolution de la sociologie des Français de l'étranger. Ces nouveaux Français de l'étranger ne trouvent pas toujours à la CFE une offre abordable correspondant à leurs besoins. En simplifiant l'offre tarifaire de la CFE en matière d'assurance maladie volontaire, en permettant un niveau de prise en charge clair et lisible en fonction du pays où les soins seront prodigués et en supprimant la condition de nationalité pour être adhérent, la présente proposition de loi répond de manière concrète à ces nouvelles formes et à ces nouveaux parcours de l'expatriation. Nous pouvons tous nous en réjouir. Si je salue le travail réalisé par la commission, je déplore néanmoins que l'élargissement du collège électoral procédant à l'élection du conseil d'administration ne figure pas dans le texte issu des travaux de la commission.

Ce collège électoral est anachronique étant donné que la réforme de la représentation des Français de l'étranger, introduite par la loi du 22 juillet 2013, a instauré 443 conseillers consulaires et a réduit à 90 le nombre des conseillers de l'Assemblée des Français de l'étranger. Néanmoins, je peux comprendre les arguments évoqués par le rapporteur et certains de mes collègues, le Gouvernement ayant récemment annoncé l'ouverture d'une réflexion sur la représentation des Français établis hors de France. Je compte donc sur le Gouvernement pour faire sorte que la représentation des assurés au sein du conseil d'administration de la Caisse fasse partie intégrante de cette réflexion. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, afin de moderniser le fonctionnement de ce formidable outil qu'est la CFE et de la faire pleinement entrer dans le XXI siècle, je vous invite à voter cette proposition de loi.

Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la Caisse des Français de l'étranger a quarante ans. Le bel âge, me direz-vous ! Je ne saurais dire le contraire, c'est le mien ! Pour autant, c'est aussi celui des remises en question, des tournants à prendre, des réorientations. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui répond à cette nécessité. Le texte que nous soumet la commission des affaires sociales n'a plus rien à voir avec la mouture initiale, et c'est heureux, car celle-ci était obsolète.

Qu'il me soit aussi permis de rendre hommage à notre ancien collègue Jean-Pierre Cantegrit, qui a fortement contribué au développement de la CFE, en présidant son conseil d'administration sans interruption depuis l'origine jusqu'en 2015. Sous son impulsion, la CFE, créée initialement essentiellement pour répondre aux besoins des entreprises qui expatriaient des cadres, a accompagné l'expansion des entreprises à l'international dans le cadre de la mondialisation, mais a également élargi son champ d'intervention à toutes les catégories de Français qui faisaient le choix de s'expatrier pour diverses raisons, qu'il s'agisse de jeunes à la recherche d'un emploi, de retraités, d'entrepreneurs ou autres. Ce modèle, qui transpose notre système de protection sociale à l'étranger, en particulier dans le champ de l'assurance santé, a trouvé progressivement ses limites pour diverses raisons diminution de l'expatriation classique du fait que les entreprises recrutent de plus en plus localement ; faible attractivité vis-à-vis des jeunes, en raison de tarifs peu compétitifs ; grilles tarifaires par statut et donc inadaptées ; modalités de prise en charge des soins peu lisibles ; difficultés à disposer d'un réseau de soins permettant d'offrir le tiers payant. Et cela s'est traduit par un recul du nombre des adhésions à la CFE, porteur à terme d'une dégradation prévisible de finances encore provisoirement saines. C'est dans ce contexte que le conseil d'administration, renouvelé en 2015, a porté Alain-Pierre Mignon à sa tête. Ce dernier est non seulement un élu des Français de l'étranger, mais aussi un chef d'entreprise dynamique et créatif, qui a mis son énergie, avec la nouvelle direction, à concevoir une stratégie dans laquelle s'inscrivent des projets visant à renforcer la protection sociale des Français établis hors de France. La mise en oeuvre de ces projets ambitieux rend nécessaire l'adaptation de la législation applicable à la CFE, et tel est l'objet de notre discussion aujourd'hui. Les clients de la CFE y adhèrent en étant rattachés à un statut : salariés, non-salariés, étudiants, retraités, inactifs. Difficile à gérer, avec des niveaux de cotisations correspondant aux ressources des assurés presque invérifiables, ce système détourne une partie des Français de l'étranger de la CFE au bénéfice d'assureurs privés. C'est dans ce contexte que la Caisse a décidé de moderniser ses grilles tarifaires, qui seront dorénavant assises sur l'âge et la composition de la famille de l'assuré. C'est un progrès considérable et une réelle simplification. Cela renforce l'attractivité de la CFE et la lisibilité des cotisations. L'innovation de la réforme qu'il nous est proposé de voter réside dans le fait non pas qu'elle fixe les nouvelles règles que la Caisse souhaite mettre en oeuvre et que nous soutenons, mais qu'elle donne au conseil d'administration de la CFE la possibilité d'adapter son dispositif tarifaire et les modalités de prise en charge des soins, dans un souci de coller plus fortement aux besoins des Français de l'étranger. Cette souplesse conférée au conseil d'administration interviendra bien entendu sous le contrôle des pouvoirs publics. Cela ne remet pas en cause le statut de caisse de sécurité sociale de base. En revanche, la loi permettra à la CFE de conclure des partenariats avec des assureurs complémentaires pour offrir à ses clients une prise en charge complète des soins qu'ils engagent. Les Français établis hors de France sont les meilleurs pour faire une analyse comparative des fonctionnements, ce qu'on appelle le « parangonnage ». Faisons-leur confiance pour savoir s'adapter et garder une caisse des Français de l'étranger performante et efficace En votant ce texte, nous améliorerons l'accès de nos compatriotes à une protection sociale française de qualité. Parce que le temps presse, que des mois de navette parlementaire feraient perdre un temps précieux à une réforme qu'il nous faut engager le plus rapidement possible, j'espère que nous trouverons une voie consensuelle

Je m'attacherai au volet principal de notre proposition de loi, à savoir celui de la tarification. La CFE couvre aujourd'hui 190 000 adhérents. Il semblerait que la Caisse ne soit malheureusement plus en mesure de fournir des réponses adaptées aux enjeux d'une couverture volontaire de qualité accessible au plus grand nombre, notamment pour la troisième catégorie, qui regroupe les assurés les plus vulnérables, lesquels ne bénéficient pas d'un régime de soins efficace dans leur pays de résidence. C'est pourquoi nous avons souhaité introduire un nouveau régime de cotisation simplifiée : la cotisation volontaire pour la couverture des frais de santé de nos compatriotes à l'étranger serait déterminée en fonction de leur tranche d'âge et de leur composition familiale. L'offre tarifaire n'est plus adaptée à la mobilité de nos compatriotes, avec plus de 600 tarifs qui entravent aujourd'hui l'amélioration des performances de la Caisse. Ainsi, notre texte prévoit une offre de prise en charge claire et lisible en fonction du pays de résidence où les soins sont prodigués, afin de parvenir au meilleur niveau de prise en charge. Il faut avoir à l'esprit que la mobilité attire principalement nos compatriotes se situant dans la tranche d'âge 20-45 ans. Leur départ de l'Hexagone est souvent lié à leurs études ou à leur plan de carrière. Or il apparaît que les tarifs pratiqués par la Caisse sont trop élevés pour ceux qui ne sont pas pris en charge par leurs entreprises, la majorité d'entre eux. Beaucoup, ensuite, s'installent dans le temps et fondent souvent une famille : leur partenaire n'adopte pas forcément la nationalité française, alors que les enfants, eux, sont français. Il nous semble donc normal que toute la famille puisse adhérer à la Caisse. La suppression de la condition de nationalité française pour l'adhésion nous paraît par conséquent justifiée, afin d'éviter toute discrimination. Néanmoins, il faut admettre que les nouveaux produits sont de nature à résorber les tarifs trop élevés. Je pense à l'assurance JeunExpat Santé, avec une cotisation de 49 euros mensuels pour les jeunes de 18 à 29 ans. Je veux aussi saluer une autre offre « Produit France », qui permet aux assurés d'opter pour un remboursement des soins réalisés uniquement en France, réduisant ainsi leurs cotisations. La majorité La majorité des jeunes Français partant à l'étranger n'a aucune couverture sociale ou celle-ci est trop souvent limitée aux premiers mois de leur expatriation. Ces mesures devraient les inciter à s'assurer grâce à des tarifs plus abordables.

Nous avons également souhaité introduire des avancées sociales, comme la suppression de l'exigence d'un montant minimal pour le versement des cotisations dues par les retraités, la fin de l'exigence du délai maximal au cours duquel l'intéressé peut demander son adhésion à l'une des assurances volontaires et, enfin, une couverture intégrale des frais relatifs aux risques et aux conséquences de la maternité. En outre, nous proposons un plafonnement de l'augmentation des cotisations à 50 % sur dix ans. Ces améliorations sont de nature à rendre efficace le modèle économique actuel, qui ne permettait plus de répondre à toutes les attentes de ceux qui n'ont aucune couverture sociale dans leur pays de résidence et de ceux qui recherchent principalement une couverture complémentaire en cas d'hospitalisation sur leur lieu d'habitation. Dans cette proposition de loi, mes collègues et moi-même nous sommes attachés- je rends hommage à l'excellent travail du président et des administrateurs de la Caisse, ainsi que du rapporteur, Yves Daudigny -à rendre la CFE plus attractive, plus accessible et, surtout, ouverte à tous. Mes chers collègues, au regard de l'ensemble des améliorations proposées quant à la politique tarifaire de la Caisse des Français de l'étranger, au coeur du présent texte, je vous invite à voter en faveur de la proposition

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 1 met en conformité le droit applicable à la CFE avec le droit communautaire, reprenant les recommandations de l'IGAS. Comme l'a dit mon collègue Olivier Henno lors de la discussion générale, j'étais intervenu en 2015 contre la proposition de loi réformant la gouvernance de la CFE. de mes collègues de la majorité sénatoriale, nous avions préféré attendre les conclusions de l'IGAS. Les différentes interventions dans le cadre de la discussion générale permettent de constater que le texte que nous examinons aujourd'hui est arrivé à maturité. En atteste, par exemple, l'élargissement des possibilités d'adhésion aux citoyens européens, prévu par l'article 1. En tant que représentant des Français établis hors de France, je suis ravi que la CFE ait pu être impliquée dans la rédaction de ce texte et que son président, Alain-Pierre Mignon, soit satisfait du résultat.

qui a permis à la commission d'amender significativement le texte initial, aboutissant à un consensus. La Caisse des Français de l'étranger est une caisse de sécurité sociale qui a mis un point d'honneur à équilibrer ses comptes en toutes circonstances, alors qu'elle évolue dans un contexte ultraconcurrentiel. Cela mérite d'être salué, et je remercie mes collègues Jacky Deromedi et Ronan Le Gleut d'avoir rappelé le rôle joué par l'ancien sénateur Jean-Pierre Cantegrit. La CFE est un outil très précieux non seulement pour nos compatriotes qui y font appel à l'étranger, mais aussi pour les entreprises qui ont besoin d'une couverture sociale pour leurs collaborateurs expatriés, ce qui favorise notre commerce extérieur.

Je lève le gage,

Merci